Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

L'annulation du salon de l'agriculture pour cause de pandémie nous oblige, nous, parlementaires, à relayer la détresse du monde rural. Alors que 2020 est une année record en matière de bénéfices pour la grande distribution, alors que les négociations commerciales ont été difficiles et ne se sont conclues que dans la nuit de lundi à mardi, les revenus des agriculteurs sont au plus bas. Comment se fait-il que l'obligation contractuelle faisant référence aux coûts de production, pourtant prévue par la loi, ne soit pas proposée aux producteurs et que les entreprises de transformation n'obtiennent pas de la grande distribution un accord à cette hauteur ? Cette situation n'est ni morale, ni acceptable, ni justifiable. Comment comptez-vous y remédier ?

J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que le Premier ministre se rendra dans les prochains jours auprès de nos éleveurs pour leur témoigner très concrètement la reconnaissance que leur doit notre gouvernement. C'est obscène !

qui doit proposer des pistes d'amélioration. Vous le savez, la transparence est la clé pour surmonter l'opposition entre distributeurs et industriels. Nous continuons à mener à bien l'application de la loi Égalim. Bruno Le Maire intensifie et démultiplie les contrôles pour qu'elle soit appliquée de manière effective. Par ailleurs, nous renforçons la médiation, dont nous savons qu'elle est indispensable. Enfin, nous avons lancé une adresse de signalement pour mobiliser les consommateurs et lutter contre des prix trop bas

La parole est à Mme Christine Herzog, pour le groupe Union Centriste.

Hier matin, à minuit, pour la seconde fois en moins d'un an, le gouvernement fédéral d'Angela Merkel a mis fin à soixante ans de relations transfrontalières entre le département de la Moselle et ses deux allemands voisins de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat. Ces ont manifesté leur mécontentement devant cette rupture brutale des accords et traités relatifs à la libre circulation des personnes et des marchandises. c'est un taux d'incidence trop élevé de la circulation du covid-19 et de ses variants en Moselle. Or c'est précisément de ce point de vue que la prise de décision allemande pose problème. Tout d'abord, il a été constaté et relevé que les allemands dépistaient quatre fois moins de personnes que les départements français. Et pour cause,

les conséquences les plus dures de ce classement. Je rappelle que ce classement a abouti automatiquement, avec les voisins autrichien et tchèque de l'Allemagne, à une fermeture complète des frontières. C'est cette situation que nous avons voulu éviter pour la Moselle, compte tenu de la réalité que vous avez rappelée, notamment pour les 16 000 travailleurs qui, quotidiennement, ont besoin de franchir la frontière pour exercer leur activité professionnelle. Nous avons pu contenir l'impact de ce classement

vous persistez dans votre obstination à aggraver la précarité des plus fragiles dans notre pays. Vous annoncez ainsi vouloir faire plus de 1,3 milliard d'euros d'économies sur le dos des demandeurs d'emploi. Oserai-je vous rappeler qu'ils ne sont pas responsables de leur situation ? Depuis des mois, en pleine crise sanitaire, les plans de licenciement se multiplient partout dans notre pays. Face à cette crise sociale qui s'aggrave, votre réponse consiste à repousser d'un an le bonus-malus pour les entreprises, imposer dès le 1 juillet prochain une baisse de 20 % des indemnités journalières à plus de 830 000 demandeurs d'emploi. On est finalement bien loin du « en même temps » de 2017 Depuis plusieurs mois, la pauvreté s'accroît dans notre pays. Les Restos du coeur, le Secours populaire, le Secours catholique nous alertent quotidiennement : les files d'attente s'allongent devant les distributions alimentaires, semaine après semaine.

sans surprise, nous ne sommes pas d'accord sur la réforme de l'assurance chômage, mais je ne peux pas laisser dire que le Gouvernement n'agit pas massivement pour lutter contre la précarité. Je vous rappelle que nous avons prolongé les droits des demandeurs d'emploi depuis le mois de novembre dernier en mobilisant plus de 1,5 milliard d'euros.

Ce sont plus de 460 000 demandeurs d'emploi qui bénéficient de cette aide, pour laquelle nous mobilisons 1,2 milliard d'euros. Je rappelle en outre que, pour lutter contre la précarité, nous utilisons l'activité partielle, ... Ce sont des acquis sociaux 9 millions de salariés au plus fort de la crise, et encore 2 millions au mois de janvier dernier. Pour ce qui est de la réforme de l'assurance chômage, le Gouvernement

pendant cette crise sanitaire que personne n'a souhaitée. Oui, au titre de ces mesures d'urgence, nous avons protégé l'activité économique, les femmes et les hommes qui, au quotidien, continuent de travailler. C'est bien normal et ce n'est pas le moment de se dire merci ! Ce que vous proposez, c'est d'aggraver, dès le 1 juillet prochain, la situation de ces femmes et de ces hommes qui aujourd'hui perdent leur emploi. Madame la ministre, vous avez déclaré, voilà peu, que vous étiez une femme de gauche, attachée à la justice sociale. La réforme que vous proposez n'est pas une réforme de gauche. Une réforme de gauche, c'est tirer les droits vers le haut, pas vers le bas

Ma question vise à vous demander un bilan des premières remontées de la concertation, qui était déjà largement engagée et qui s'approfondit. Des maires ont fait parvenir des suggestions intéressantes et utiles.

Les élus de tous bords, y compris du sien, partout en France, se sont d'ailleurs réfugiés dans un silence assourdissant, dont je sais qu'il est en réalité réprobateur. Sénateur de Paris, j'ai été très choqué- je le dis -que n'aient été consultés ni les maires d'arrondissement ni les élus franciliens, comme si Paris était une citadelle et comme si le virus allait s'arrêter à ses portes.

Le taux d'incidence remonte partout, mais la situation est particulièrement préoccupante à Mayotte, à La Réunion, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en PACA. Nous suivons cela de très près avec Olivier Véran. Nous déployons à cette fin un arsenal de mesures visant à briser la dynamique épidémique : suivi des cas contacts, respect de l'isolement des patients et des cas contacts. Nous accompagnons les collectivités touchées par des mesures de gestion dédiées.

rester collectivement vigilants. Cette vigilance s'exerce au quotidien par le respect des gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, le recours au télétravail quand cela est possible. Nos concitoyens ont consenti à de nombreux sacrifices qui ne sauraient être balayés sur l'autel d'enjeux partisans. Dans un esprit de concorde, nous tenons à consulter et à associer les collectivités concernées dans l'élaboration des réponses les plus adéquates en phase avec les dynamiques territoriales.

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pour la première fois dans notre histoire récente, un ancien Président de la République a été condamné à trois années d'emprisonnement pour « corruption active » et « trafic d'influence » par le tribunal correctionnel.

Lorsque le ministre de l'intérieur s'exprime face caméra en déplacement officiel, le propos qu'il tient n'est pas un propos privé : c'est la position du Gouvernement. Oui ! Monsieur le Premier ministre, ma question est simple : partagez-vous les propos de votre ministre de l'intérieur ? Considérez-vous qu'ils soient compatibles avec sa fonction ?

Marie-Pierre de La Gontrie, vous êtes une spécialiste des questions institutionnelles et des questions judiciaires. Vous savez donc qu'en tant que membre du Gouvernement je n'ai pas de commentaire à faire sur une décision de justice. C'est déjà fait ! Il y a une séparation des pouvoirs et un État de droit.

Monsieur le Premier ministre, votre silence est éloquent. Vous avez souhaité ne pas répondre et, finalement, nous ne saurons pas si vous partagez ou non les propos du ministre de l'intérieur. Pour ma part,

de la loi et l'indépendance de l'autorité judiciaire. Comment ne pas voir l'effet dévastateur de l'expression publique d'un soutien amical adressé par le patron des policiers à une personne lourdement condamnée pour des manquements à la probité ? Monsieur le Premier ministre, nul ne peut se réjouir de voir un ancien Président de la République condamné pour corruption, mais tous nous devrions nous réjouir d'avoir une justice qui s'applique à tous, puissants ou misérables.

L'État et la région Occitanie travaillent actuellement à un protocole relatif aux lignes de desserte fine du territoire de ladite région. Cet accord doit permettre de matérialiser les engagements respectifs de l'État, de la SNCF et de la région. vous avez souhaité exclure les lignes de l'Aubrac et des Cévennes de ce protocole afin de les traiter dans un accord interrégional ultérieur associant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le souhait d'un tel report renforce les inquiétudes sur les intentions du Gouvernement concernant la ligne de l'Aubrac.

d'abord, parce qu'elle relie, comme le Cévenol, la Lozère à notre capitale. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas des sous-citoyens : comme tous les Français, nous avons le droit à des infrastructures qui nous permettent de rejoindre Paris en un temps raisonnable. ensuite, parce que la ligne de l'Aubrac achemine de nombreux lycéens et étudiants vers leur lieu de formation et assure le fonctionnement et la viabilité de l'une des dernières usines sidérurgiques françaises, une entreprise innovante dans le domaine des aciers électriques haut de gamme. enfin, parce qu'elle permet chaque année à des centaines de touristes d'accéder à l'Aubrac. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, ma question est plurielle. Où en est cette convention ? Que contiendra-t-elle ? Quels sont les engagements de l'État et de la SNCF pour satisfaire les besoins urgents d'investissement en matière de régénération de cette ligne ?

vous m'interrogez sur la desserte du Massif central, ce qui me permet de revenir brièvement sur la politique du Gouvernement en matière ferroviaire. Comme vous le savez, en 2017, nous avons concentré notre action sur les lignes du quotidien en suspendant pour un temps les grands projets, de manière à assainir la situation financière de la SNCF, avec 35 milliards d'euros de dette reprise, à réinvestir massivement sur le réseau ferroviaire- plus de 3 milliards d'euros par an -et à engager le sauvetage des petites lignes ferroviaires en lien avec les régions, pour un volume de 6,5 milliards d'euros

Au-delà d'un engagement financier ponctuel, ma question porte bien sur l'engagement à long terme de l'État. Au-delà du Grand Paris, il y a la France. Chaque territoire mérite l'investissement de l'État. La parole est à M. Ronan Dantec, pour le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires.

du Président de la République d'une déclinaison « sans filtre » des travaux de la Convention citoyenne, le Gouvernement a décidé de les repasser à la moulinette, hachant menu, très menu, l'ambition initiale et le mandat donné aux 150 citoyens Ainsi, alors que nous savons qu'il faut dix ans pour que nos décisions politiques aboutissent à des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre, vous décidez aujourd'hui que la France n'honorera en en 2030 ni l'accord de Paris ni l'objectif européen de réduction de 55 % des émissions de CO2, objectif que vous avez pourtant soutenu lors du Conseil européen du 11 décembre dernier. et environnemental (CESE), le Conseil d'État et le Haut Conseil pour le climat pointent tous l'insuffisance du projet de loi et ses incohérences ? Le Haut Conseil pour le climat conclut même que le texte permettra au mieux 20 % de réduction des émissions en 2030. Ma question est donc simple. Au mois de novembre prochain, la COP26 sera consacrée au rehaussement de l'ambition. Gouvernement compte-t-il assumer, à Glasgow, cet adieu français à l'accord de Paris, que nous avions pourtant promu il y a six ans par une mobilisation exceptionnelle de notre diplomatie ?

Je tiens d'abord à rappeler le caractère totalement inédit de cette démocratie participative, qui a permis, sous l'impulsion du Président de la République, à 150 citoyens de se

essentielle. Nous avons longuement et continûment échangé avec les citoyens. Ceux-ci ont rendu un jugement sur l'action du Gouvernement, en toute indépendance. Il appartient maintenant au Parlement de se saisir du texte et de remplir sa fonction, au nom du peuple français.

par voie réglementaire et 14 sont intégrées dans le projet de loi de la Convention citoyenne. Nous avons pu ainsi avancer sur des sujets majeurs. Je pense notamment à la conversion du parc automobile, qui aura des impacts et des résultats très significatifs en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, à la création de trente-cinq zones à faibles émissions, qui permettent là aussi de lutter contre la pollution de l'air dans les zones les plus densément peuplées, ou encore à la multiplication du plan Vélo que vous appelez de vos voeux, monsieur le sénateur. Notre vision est simple. Nous agissons en complémentarité des modes de transport et non en concurrence. Nous organisons l'équité entre les territoires. Nous mettons en oeuvre des transitions industrielles dans un souci de justice sociale, car vous savez que certains secteurs subissent des mutations extrêmement profondes.

consultés. Ils représentent pourtant 79 % des effectifs ... En rapport avec la directive européenne de 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, cette missive indique que les sapeurs-pompiers volontaires pourraient être considérés comme supplétifs de fait, risquant donc d'être assimilés à des professionnels. Cela irait à l'encontre du refus de transposer la directive aux sapeurs-pompiers volontaires, position qui est défendue depuis 2003 par tous les parlementaires et tous les gouvernements. La loi du 20 juillet 2011 est très précise et indique que « l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel ». En 2019,

la désorganisation du fonctionnement des SDIS, la dégradation des délais des secours et la disparition progressive de ce service public solidaire.

comme vous le pointez justement dans votre question, le ministère de l'intérieur a bien adressé une communication aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours au mois de novembre 2020, à de la réponse de la Commission européenne sur la question de la directive européenne du temps de travail, la DETT. Il s'agit bien d'un message pour leur annoncer cette concertation. Il existe aujourd'hui un consensus partagé par une très grande majorité des parties prenantes sur la nécessité d'adapter notre modèle actuel de volontariat. Ce de remettre en cause son mode de fonctionnement, qui a largement fait ses preuves- vous l'avez très bien rappelé -tant au quotidien que dans les crises- je salue le travail des sapeurs-pompiers volontaires partout en France -, mais bien de veiller à encadrer certains points qui pourraient notamment risquer de conduire à des décisions de justice contraires au principe de l'engagement citoyen que nous défendons collectivement ici. C'est donc bien sous le sceau de la transparence et de la concertation que le ministère de l'intérieur a voulu engager ces travaux, qui doivent nous permettre de trouver des solutions aux problématiques soulevées par la directive européenne de 2003 concernant certains aspects

La réflexion qui vient de s'engager doit pouvoir permettre, en liaison étroite avec les SDIS ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs et partenaires, de disposer de leurs analyses sur ces problématiques, mais aussi de leurs propositions. Monsieur le sénateur, je tiens à vous dire ici, au nom du ministère de l'intérieur, que nos objectifs sont clairs : maintenir une organisation efficace des SDIS sans perdre de potentiel opérationnel et proposer une solution concertée et soutenue par l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, qui ne porterait pas atteinte à notre modèle de volontariat,

Les Républicains. Madame la ministre de la cohésion des territoires, comme moi, vous entendez les préoccupations et les inquiétudes grandissantes des collectivités locales, plus particulièrement des communes et des intercommunalités, qui sont fortement mobilisées,

imputables à la crise sanitaire. Par ailleurs, 25 % des intercommunalités jugent aujourd'hui que leur situation financière est dégradée. Les collectivités concernées demandent et méritent toute notre attention. Madame la ministre, devant l'hétérogénéité des situations dans nos territoires, quels plans d'action le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre pour soutenir les collectivités, leur permettre de préparer la sortie de crise et de préserver les investissements locaux ?

comme vous le savez, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures de soutien aux collectivités territoriales, dont les finances ont été très touchées par la crise que nous traversons.

des recettes de fonctionnement et une hausse de 0,2 % des dépenses de fonctionnement, toutes collectivités territoriales confondues. Ainsi, même si l'épargne brute diminue si l'épargne brute diminue de 3,7 milliards d'euros, elle se maintient au même niveau qu'en 2018 et bien au-dessus des niveaux des années précédentes. Cette tendance souligne que les budgets locaux sont

(RSA) de plus, 230 000 chômeurs de plus : est-ce là une opportunité pour une relance de la réforme de l'assurance chômage ? C'est anachronique et provocant ! Vous annoncez votre réforme pour l'été 2021, en pleine tempête économique, alors que le recours au chômage est plus que jamais un instrument d'équilibre et de justice.

Il faudra désormais avoir travaillé six mois sur vingt-quatre au lieu de quatre mois sur vingt-huit pour accéder à une allocation, alors que tant de nos entreprises, surtout les plus petites, sont en difficulté et peinent à maintenir leurs emplois. C'est sur les plus fragiles, les précaires, que vous faites peser vos objectifs d'économies, en diminuant leurs droits et en estimant qu'ils font le choix du chômage ! C'est faux ! Ils le subissent ! Les plus affectés par l'impact de la crise touchent en moyenne 1 300 euros ! Est-ce sur eux qu'il faut réaliser vos économies ? Les Français sont inquiets. La pauvreté s'accroît de manière dramatique depuis l'arrivée de la covid, malgré la solidarité nationale. Alors qu'il faudrait créer les conditions de la confiance, vous ajoutez à l'inquiétude profonde de la population des sentiments d'injustice, d'incertitude et de détresse. Tous les partenaires sociaux sont contre. C'est cela, la gauche ! Nous sommes nombreux à vous demander d'abroger ce projet de réforme conçu en 2019, dans un tout autre contexte, et inadapté en temps de crise de l'aveu même de l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Allez-vous poursuivre malgré ces alertes, au risque d'une véritable casse sociale ?

La réforme que j'ai présentée hier aux partenaires sociaux est le fruit de six mois d'échanges ininterrompus au cours desquels j'ai écouté les observations, les propositions des uns et des autres. Cette réforme repose sur deux principes : lutter contre la précarité et assurer plus d'équité dans le calcul des allocations chômage. La réforme met en place un système de bonus-malus qui encourage les entreprises vertueuses en termes d'emploi et qui dissuade les entreprises qui recourent excessivement aux contrats courts. Je pense que nous pourrions nous retrouver sur cette mesure. Contrairement à ce que j'entends dire parfois, la réforme ne réduit pas les droits des allocataires. Le montant total des allocations est strictement conservé, ce qui signifie que, si l'allocation mensuelle baisse pendant un mois donné, elle est servie plus longtemps. Par ailleurs, la concertation nous a conduits à mettre en place un plancher pour éviter des allocations trop basses. Je rappelle également que, depuis le début de la crise, nous agissons massivement contre la précarité par la mise en place de l'activité partielle, en prolongeant, quand c'est nécessaire, les droits des demandeurs d'emploi et en mettant en place une aide exceptionnelle pour les travailleurs les plus précaires

La moitié des transactions du marché des actions ont migré vers l'Union européenne. Contre toute attente, après quatre siècles, Amsterdam est devenue la première place financière européenne, devant Londres. Paris maintient sa troisième place, en légère progression, mais loin derrière, près deux tiers des transactions de la Bourse de Londres. Il est vrai que les gouvernements français ont fait pendant longtemps la promotion de la fiscalité néerlandaise, en plaçant les participations de l'État sur la place néerlandaise, à La Il est vrai aussi que cela a inspiré des groupes nationaux tels que le groupe Vivendi, qui annonce la capitalisation de sa filiale Universal à La Haye dans quelques mois.

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le sénateur Dominati, vous posez une question relative à l'attractivité de la place et de la Bourse de Paris. C'est en effet un sujet essentiel sur lequel le Gouvernement est mobilisé depuis 2017. C'est un peu tard ! Non, ce n'est pas trop tard ! La France conduit un vaste programme de réformes visant à renforcer la place des services financiers

ainsi que pour les applications relatives à la. Vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, depuis 2019, Paris a cherché et a réussi à attirer des acteurs financiers internationaux. Je pense à la relocalisation des plateformes de négociation de Goldman Sachs et d'Acquis Exchange. Je pense aussi à l'ouverture du nouveau bureau de Citadel et à la création des filiales européennes de Chubb et de Bank of America, qui sont autant d'exemples illustrant concrètement l'attractivité croissante de la place. Paris est ainsi le seul centre financier continental à avoir réussi à capter l'ensemble de l'écosystème des services financiers. Monsieur le sénateur, vous savez que, depuis le 1 janvier 2021 et à la fin de la période de transition du Brexit, les actions d'entreprises de l'Union échangées en euros ne peuvent plus être échangées sur les plateformes boursières du Royaume-Uni à qui la Commission européenne a décidé de ne pas octroyer d'équivalence. Ce mouvement important de rapatriement des échanges d'actions dans l'Union européenne a conduit à la relocalisation dans des principales plateformes internationales d'échanges d'actions. Paris, aux côtés d'Amsterdam que vous mentionnez, en a été l'un des deux principaux bénéficiaires en attirant sept plateformes anglo-saxonnes, notamment la

ne s'intéresse pas à la région parisienne et au Grand Paris. C'est le premier gouvernement sous la V République qui traite aussi mal la région capitale !

En 2018, la « ferme France » a conservé son statut de première puissance agricole européenne, avec une production estimée à 73 milliards d'euros et une contribution au PIB de 6,7 %. Ces chiffres démontrent la compétitivité et la performance de l'agriculture française. Elle est la meilleure du monde en termes qualitatifs, nutritionnels et environnementaux En des temps normaux, nous devrions rencontrer, à cette période de l'année, les agriculteurs de nos territoires au salon de l'agriculture, à la porte de Versailles. À défaut, cette année sont proposées des journées sur tout le territoire ! Les années suivantes ne ressembleront pas à 2021, et c'est heureux. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe Union Centriste, nous demandons simplement et symboliquement la création d'une journée nationale de l'agriculture.

ou les dégâts de la grippe aviaire, pour n'en citer que quelques-unes. Il s'agit bien au contraire de valoriser les métiers de l'agriculture ! Cette journée permettra aux acteurs de la filière de mettre en valeur la spécificité des territoires et les nouvelles techniques plus durables. Elle doit permettre aux citoyens de connaître les femmes et les hommes passionnés qui nourrissent la population ! Il s'agira d'un geste fort qui sortira le secteur agricole de son sentiment de découragement et marquera la considération que l'ensemble du pays

il faut aussi faire connaître nos agriculteurs et leur métier. C'est la raison pour laquelle mon collègue ministre de l'agriculture m'indique plusieurs éléments qui, je le crois, répondront à votre suggestion et proposition. D'abord, le Centre national des expositions et concours agricoles organisera au printemps prochain la semaine française de l'agriculture, avec des échanges et des conférences. Ensuite, les journées nationales de l'agriculture se dérouleront au mois de juin prochain. Elles permettront aux Français, comme vous le souhaitez, de visiter des exploitations et de saisir la réalité du métier

Ma question s'adresse à Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Madame la ministre, vous avez fait le choix de poursuivre la discussion avec les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage et nous ne pouvons que vous en féliciter. La question de la temporalité et des réformes successives sur ce dossier se pose. La crise économique ne gomme pas le contexte dans lequel nous nous trouvons. Le contexte

tend à rendre le service public de l'emploi plus dépendant de la conjoncture économique, ce qui dessine des perspectives financières extrêmement incertaines pour Pôle emploi en 2022. Nous vous tendions la main en proposant que le document de cadrage adressé aux partenaires sociaux sur ce sujet fasse l'objet d'une discussion au Parlement, ce qui a été balayé d'un revers de manche par le gouvernement précédent. Il s'agit enfin incertain sur l'état réel du marché du travail et de certains secteurs. Mes questions sont donc au nombre de trois. Pensez-vous que les discussions d'hier vont renouer les liens et faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage ? Ne pensez-vous pas que, pour cette réforme, il faille accepter de travailler davantage avec le Parlement, les régions et les départements, avant la publication d'un décret qui gravera dans le marbre les futures règles d'indemnisation des années à venir ? Ne faut-il pas, au regard de la conjoncture, envisager des solutions à géométrie variable selon les branches ou les secteurs géographiques, qui seront sans doute touchés de façon différenciée les uns des autres ?

comme vous, je suis attachée au dialogue social et je suis convaincue que les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel depuis le début de la crise. C'est la raison pour laquelle, au cours des six derniers mois, j'ai écouté les propositions et les observations formulées par les C'est ainsi que nous avons construit la réforme que j'ai présentée hier. Par exemple, en réponse aux observations des organisations syndicales, nous avons fait le choix de décaler au 1 juillet prochain la mise en oeuvre de cette réforme,

une considération de bon sens, à savoir que les paramètres de l'assurance chômage doivent pouvoir s'adapter pour tenir compte de la situation du marché du travail. En outre, vous l'avez vu, nous avons instauré un plancher pour éviter les allocations trop basses, comme les organisations syndicales nous le demandaient. ailleurs, pour répondre également aux inquiétudes des organisations patronales, nous avons aménagé le dispositif de bonus-malus, afin que les périodes « atypiques »- l'année 2020 et le début de l'année 2021 -n'entrent pas en compte dans le calcul de ce bonus-malus et que les secteurs les plus affectés par la crise ne soient pas concernés. C'est cette écoute permanente des organisations patronales et syndicales qui nous a permis d'élaborer la réforme présentée hier. Par ailleurs, nous devons ouvrir, avec les partenaires sociaux,

Ces sommes portent en elles toute l'iniquité de cette crise : sans surprise, 70 % du surcroît de l'épargne est le fait des 20 % des ménages les plus riches en France. L'argent n'est pas fait pour être entassé, il est fait pour circuler. Les tergiversations du Gouvernement sur la question coûtent cher à la France ! En matière de libéralisation de l'épargne, la confiance est cardinale. En ce sens, les atermoiements sur la politique vaccinale ne sont malheureusement pas de nature à restaurer cette confiance, dont nous avons tant besoin. Je n'appelle pas à toucher à l'épargne de précaution accumulée par nos concitoyens les plus modestes, mais je vous demande de mettre à contribution ceux pour qui la crise a permis cette accumulation. Rétablir l'ISF pour contribuer à l'effort de solidarité C'est non ! Taxer l'épargne des plus aisés pour relancer l'économie ? Encore non ! En refusant cela, vous actez votre renoncement à faire contribuer ceux pour qui la crise a été synonyme d'enrichissement. Une mobilisation par l'impôt permettrait d'instaurer une répartition plus égalitaire de l'effort de relance. de relance. Le virus se propage sur un terrain déjà miné par les inégalités ; celles-ci n'ont cessé de se creuser dans des proportions inédites. Comment comptez-vous mobiliser ce fonds de guerre, thésaurisé par les citoyens les plus aisés, afin qu'un embryon de justice fiscale puisse enfin voir le jour dans votre quinquennat ? Il vous reste encore un an. Rien n'est jamais trop tard ... La parole est La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le sénateur Cozic, vous m'interrogez sur le fléchage de l'épargne vers la relance de l'économie, sujet sur lequel le Gouvernement est mobilisé depuis 2017.

Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, à peu près 200 milliards d'euros d'épargne sont disponibles. Vous parlez de trésor, mais c'est surtout l'argent des Français. Notre objectif est clair : que cette épargne serve au financement de l'économie réelle, de nos entreprises. C'est dans l'intérêt des épargnants- cela leur rapporte de la rentabilité, dans un contexte de taux bas -, mais aussi, voire surtout, dans celui de nos entreprises, qui ont toujours besoin de ces ressources pour investir,

permet aux épargnants d'identifier les fonds qui ciblent tout particulièrement les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres, dans les entreprises françaises, notamment dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire.

à leur épargne ; ils sont de plus en plus nombreux. Enfin, nous avons mis en oeuvre des mécanismes pour flécher l'épargne vers des entreprises à impact et nous incitons de plus en plus chaque Français à mettre

Lillibelle et Toumani, 14 ans, sont morts dans l'Essonne, lundi et mardi derniers, respectivement à Saint-Chéron et à Boussy-Saint-Antoine, deux charmantes et paisibles bourgades, à la suite d'affrontements entre jeunes. C'est l'horreur absolue Rien de bien nouveau », me direz-vous, puisque l'amnésie collective ou le parfum de bonne conscience nous font par exemple passer sous silence le meurtre du jeune Romuald, 14 ans lui aussi, lâchement abattu en pleine rue, à Courcouronnes, le 8 novembre 2000, victime gratuite d'une vieille histoire d'impayé entre deux familles sur fond de rivalités entre quartiers. Notre pays regorge de sociologues éminemment compétents. Nous croulons sous les analyses pertinentes et détaillées du phénomène de violences en bandes, gangs ou autres tribus. Bien sûr, le sujet est extrêmement complexe ; bien sûr, la prévention ; bien sûr, l'accompagnement ... Cependant, quand répondrez-vous enfin à l'appel de détresse des élus de l'Essonne, obligés, par exemple, de quémander les crédits de leur plan de prévention spécialisée ?

calquerez-vous enfin l'évolution des effectifs de police et de gendarmerie sur la croissance démographique exponentielle d'un département comme le nôtre, ce que nous demandons en vain depuis des années

comme je le fais aujourd'hui, sur l'insuffisance des effectifs de police et de gendarmerie dans le département de l'Essonne ! C'était il y a trente-deux ans

qu'elle dure, la crise sanitaire soulève chaque jour son lot de questions, une question essentielle se pose : comment rattraper notre cap vaccinal ? accélérer la campagne de vaccination en France, je tiens à vous interroger sur les doses fantômes dont notre pays semble se priver. En effet, selon de nombreux professionnels de santé, alors que seules dix doses sont initialement prévues dans les flacons des vaccins Moderna,

Ainsi, sous réserve de certaines précautions, il serait possible de vacciner plus de personnes avec la même quantité de vaccin. Dans une commune de 4 000 habitants-

Après des tensions d'approvisionnement, on imagine aisément le gaspillage que cela représente à l'échelle nationale et le potentiel inutilisé qui pourrait profiter à cette stratégie de vaccination. de vaccination. Les autorités médicales évoluent sans cadre et risquent parfois des poursuites si elles utilisent cette onzième dose. Aussi, quelle réponse leur apporter face à ce paradoxe insupportable ? Pourquoi ne pas utiliser ces doses supplémentaires pour des patients ayant déjà été infectés par le virus et pour lesquels la Haute Autorité de santé recommande l'utilisation d'une seule dose ? La parole

C'est à cette fin que l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Moderna prévoit que chaque flacon contient dix doses. Néanmoins, afin de s'assurer dans les meilleurs délais qu'il nous soit possible d'exploiter éventuellement une onzième dose, l'État a mis, par anticipation, à disposition des établissements de santé et des centres de vaccination

La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance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

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en parvenant à un accord avec le Royaume-Uni, nous avons évité le pire,

Au moment où nous aurions besoin que l'Europe s'affirme comme un pôle de stabilité et de paix dans un monde marqué par le recul du multilatéralisme et le recours de plus en plus décomplexé à la force, notre continent s'est, en vérité, divisé et affaibli. Comme c'est trop souvent le cas, l'Europe a, d'elle-même, fait le jeu de ses concurrents et de ses adversaires. Il nous faut être lucides : aucun pays européen ne sortira gagnant du Brexit

même en l'absence de droits de douane, cet accord débouche sur le rétablissement des frontières, d'où des frictions et la désorganisation des chaînes logistiques de nos économies. Il est à craindre que la réduction des échanges ne soit plus importante que prévu et n'entraîne une réévaluation du risque économique ; les journaux rapportent quotidiennement de multiples exemples de difficultés commerciales ou industrielles que rencontrent les entreprises. Rappelons-le, le produit intérieur brut (PIB) britannique représentait 15 % du PIB de l'Union européenne. Par ailleurs, nous avons maintenant devant nous la négociation de nombreux accords sectoriels. Je ne reviens pas sur le difficile dossier de la pêche ; il semble que, pour 2021, au-delà du problème des licences, nous soyons en passe de trouver un accord pour les quotas. Toutefois, pour l'avenir, à partir du mois de juillet 2026, tout accord sur la possibilité de pêcher dans les eaux britanniques reste à écrire, donc à négocier.

tous les biens transitant entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord matérialisera une séparation commerciale. Cela ne viendra-t-il pas renforcer les courants d'opinion favorables à une réunification irlandaise ? De son côté, le parti indépendantiste écossais pourrait faire campagne en faveur d'un nouveau référendum d'indépendance, après les élections au parlement d'Écosse du printemps

Nous n'en sommes pas là, bien sûr, mais les questions irlandaise et écossaise montrent que, au-delà des difficultés économiques actuelles, les conséquences du Brexit pourraient être plus grandes encore dans le domaine politique. J'en viens au chapitre crucial de la défense et de la sécurité, pour lequel le Royaume-Uni est notre partenaire naturel en Europe. Pour ce qui concerne la relation bilatérale de défense, de défense, nous ne sommes pas trop inquiets, même si nous devons rester mobilisés pour continuer de développer le cadre des accords de Lancaster House. Il faudra continuer à faire vivre ces accords dans leurs trois dimensions : nucléaire, opérationnelle et capacitaire. Le 2 novembre dernier, nous fêtions les dix ans de ces accords. Quelques jours plus tard, le volet capacitaire connaissait une nouvelle avancée, Thales ayant eu le feu vert de la et de la Marine française pour que le programme de guerre des mines de guerre des mines entre enfin en phase de production. C'est un fait : en matière de défense, il y a une grande symétrie et de fortes synergies potentielles entre les deux ex-puissances coloniales, aujourd'hui puissances ultramarines, que sont la France et le Royaume-Uni. En revanche, nous sommes plus inquiets quant à la volonté des Britanniques de rester arrimés à la défense européenne, en dehors du cadre otanien. La réserve dont le Royaume-Uni ne s'est jamais départi en matière de politique de défense et de sécurité commune ou les déclarations récentes des responsables britanniques ne sont pas franchement de nature à nous rassurer sur ce point

Monsieur le secrétaire d'État, au-delà des postures, quelle perception avez-vous aujourd'hui de l'état d'esprit des Britanniques, en matière de défense et de sécurité européenne ? Jouent-ils simplement la montre, pour ne pas paraître en position de demandeurs ?

sur ce sujet ? Se pourrait-il qu'ils envisagent de tourner le dos à la construction de la défense européenne, alors même que leurs intérêts de sécurité sont largement les mêmes que les nôtres ? Il faudra peut-être alors que l'Union européenne assume de conquérir son autonomie stratégique avec une seule des deux principales armées d'Europe. Sans doute le Brexit ouvre-t-il à l'Allemagne de nouvelles perspectives dans ce domaine,

ainsi que l'illustre la démarche de la boussole stratégique, lancée sous la présidence allemande et que conclura la présidence française. En conclusion, je reviendrai sur les causes du Brexit, car il me semble nécessaire d'en tirer toutes les conséquences afin que, pour l'avenir, nous ne soyons plus exposés à ce type de traumatisme, qui risquerait de nous coûter bien cher, La désaffection à l'égard de l'Europe, que nous mesurons aussi en France, nous la devons tantôt à un excès de libéralisme, tantôt à un excès de bureaucratie, c'est-à-dire au sentiment mélangé d'une protection insuffisante et d'une prolifération réglementaire étouffante. Les citoyens européens ne perçoivent plus assez pourquoi nous avons fait l'Europe. Paradoxalement, la montée des périls dans le monde, jusqu'à nos frontières- je pense par exemple à la Méditerranée -, devrait redonner tout son sens à une construction européenne, qui a d'abord été conçue comme un moyen d'assurer la paix et la sécurité des Européens. Il semble que nous soyons en passe de corriger certains défauts. Désormais, face aux dégâts sociaux de la désindustrialisation, l'Europe commence à surmonter sa naïveté dans sa manière d'aborder les échanges économiques avec ses partenaires

En dépit de ses lenteurs et de ses ratés, la stratégie vaccinale européenne illustre tant cette solidarité que l'embryon d'une capacité à agir dans l'urgence. Enfin, la construction de la défense européenne et la reconquête de notre autonomie stratégique renforcent la conscience d'un destin partagé, dès lors que sont identifiées des menaces communes.

le 23 juin 2016, coup de tonnerre ! Qui imaginait alors qu'un État membre puisse quitter l'Union européenne ? C'est pourtant bel et bien arrivé ! Le Brexit est un événement inédit dans l'histoire de l'Union européenne. Ce n'est pas un événement heureux, mais cela a le mérite de rappeler que nul n'est prisonnier du projet européen. Les négociations que le Brexit a impliquées n'ont pas été un long fleuve tranquille, en raison des péripéties internes de la vie politique britannique et de la pandémie, mais elles ont également eu une vertu : celle de manifester l'unité des Vingt-Sept et de révéler le prix qu'ils accordent au marché unique, désormais clairement identifié comme l'acquis majeur de la construction européenne. Grâce à la ténacité de Michel Barnier, ces négociations se sont conclues à Noël par un accord substantiel qui satisfait les deux parties. Pourtant, comme l'a indiqué Michel Barnier lors de son audition, le 16 février dernier, c'est bien un accord « perdant-perdant car le Brexit ne profite à personne. Néanmoins, cet accord minimise les pertes. Sur l'initiative du groupe de suivi du Brexit, créé en 2016, le Sénat a adopté, voilà un an, une résolution européenne sur le mandat de négociation confié par les Vingt-Sept à Michel Barnier. Nous avons ainsi pu fixer nos lignes rouges. Au terme des négociations, Christian Cambon et moi-même avons sollicité l'organisation de ce débat en séance publique sur l'accord finalement conclu, car l'importance de celui-ci est grande pour l'Union européenne. En effet, 3,5 millions d'Européens vivent au Royaume-Uni et ce pays représente 15 % des exportations extracommunautaires. Notre résolution du mois de mars 2020 a globalement été suivie d'effets. De fait- c'était l'objectif principal, tant nos économies sont imbriquées -, l'accord de commerce et de partenariat permet la mise en place d'une zone de libre-échange entre l'Union européenne et le Royaume-Uni il garantit l'absence de quotas et de droits de douane. En contrepartie, pour prévenir tout dumping susceptible de fausser ce libre-échange, le Royaume-Uni s'engage doublement, d'une part, à ce que l'octroi des aides soit encadré par des principes communs, d'autre part, à ce que le niveau de protection réglementaire applicable dans l'Union européenne à la fin de la période de transition soit maintenu, en matière sociale et environnementale. Sur ces deux volets, si le Royaume-Uni était tenté de diverger, l'Union européenne pourra adopter des mesures compensatoires, y compris des suspensions croisées, rétablir des tarifs, voire tout remettre en cause. Cette clause dite de « non-régression » est une première dans un accord commercial et assure une concurrence loyale. ailleurs, le volet relatif à la pêche a été intégré à l'accord final, comme le demandait le Sénat. Le combat a été difficile, surtout en raison de son enjeu symbolique pour le Royaume-Uni, qui voulait retrouver sa souveraineté dans ses eaux., eaux., l'accès aux eaux britanniques est garanti pendant cinq ans et demi et nos quotas de pêche y sont certes réduits- c'était inévitable -, mais de 25 % seulement au cours de cette période. N'oublions pas que l'absence d'accord aurait privé nos pécheurs des 650 millions d'euros qu'ils pêchent chaque année en eaux britanniques. Après le 30 juin 2026, il s'agira d'une tout autre affaire : l'accès aux eaux et aux ressources reposera sur un régime de négociation annuel. En cas de remise en question des accès à l'issue de cette période, l'accord autorise les parties à adopter des mesures compensatoires. Nos répliques pourront être à la fois internes au secteur de la pêche et croisées : ainsi, Michel Barnier a fait valoir que l'accord prévoyait une clause miroir dans le secteur de l'énergie, puisque l'interconnectivité électrique- essentielle pour l'économie britannique -sera elle aussi revue dans cinq ans et demi.

du moins, en partie -, mais aussi la sécurité intérieure à travers la coopération judiciaire et policière en matière criminelle ou encore la lutte contre le blanchiment. Bien sûr, nous pouvons regretter que le Royaume-Uni se retire du programme Erasmus. Nous pouvons encore plus déplorer qu'il ait refusé d'organiser un cadre pérenne pour notre coopération en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Il faut se rendre à l'évidence : plus rien n'est comme avant. Passeports, tampons, visas, contrôle aux frontières- même pour le commerce de marchandises -sont autant de mots qui reviendront dans notre langage quotidien commun avec le Royaume-Uni. Faire respecter nos standards est un enjeu. Garantir une concurrence loyale et sécuriser les produits alimentaires sont des exigences. En matière de services, la reconnaissance mutuelle n'a plus cours, notamment pour les qualifications professionnelles. Quant aux services financiers britanniques, ils ont perdu le passeport européen et sont suspendus aux décisions d'équivalence que l'Union européenne ne prendra que si elle y a intérêt. Même sur les sujets réglés par l'accord, posons-nous encore des questions.

à se demander s'ils ne seraient pas mieux servis en arborant un pavillon britannique plutôt que français. Il s'agit, par ailleurs, de veiller aux contrôles qu'il faut désormais opérer sur nos échanges avec les Britanniques, notamment l'asymétrie des contrôles vétérinaires. Nous avons des retours d'entreprises qui bénéficient aujourd'hui de la clémence britannique. Elles craignent un retour de bâton après le 1 avril prochain. À ce titre, nous avons l'expérience douloureuse de l'embargo avec la Russie. Je m'inquiète aussi des différences de contrôles entre les États membres. L'organisation des contrôles dans les ports européens les plus concernés, du Havre jusqu'à Hambourg, n'est pas aussi rigoureuse. Certains de ces ports sont tentés de réduire les contrôles pour attirer la marchandise. Nos ports doivent s'organiser face à la concurrence des autres ports européens, d'autant que s'y ajoutera bientôt celle des ports francs annoncés par les Britanniques. surtout préoccupé par les difficultés que soulèvent les nouveaux contrôles organisés en mer d'Irlande. Le protocole irlandais annexé à l'accord de retrait a évité le pire, à savoir le rétablissement d'une frontière entre les deux Irlande. Reste que le statut hybride de l'Irlande du Nord, incluse à la fois dans le marché unique et dans le territoire douanier britannique, crée de nouvelles tensions.

y consacrera une ligne budgétaire de 5 milliards d'euros. La part qui revient à la France doit compenser l'impact du Brexit qui affecte tout spécialement notre pays, en raison de sa proximité géographique, historique et économique avec le Royaume-Uni. Nous savons que la négociation ne sera pas aisée pour partager cette enveloppe entre les Vingt-Sept. Aussi Christian Cambon et moi-même proposerons-nous bientôt au Sénat une résolution européenne pour appuyer les demandes françaises. pouvez-vous d'ores et déjà nous assurer que des critères justes et transparents présideront à la répartition des fonds obtenus entre les secteurs et les régions les plus touchés de France ? Je resituerai, pour terminer, notre débat d'aujourd'hui dans une perspective plus large, comme l'a l'a fait Christian Cambon. N'oublions pas de nous interroger sur ce qui a conduit au Brexit. Comme nous y a invités Michel Barnier, il importe de tirer les leçons du Brexit et de réfléchir ensemble à la manière de rapprocher Bruxelles des citoyens européens

presque cinq ans après le vote des Britanniques exprimant leur volonté de sortir de l'Union européenne et à l'issue d'un an de négociations difficiles entrecoupées par la crise sanitaire, un accord a enfin été trouvé. La performance mérite d'être soulignée tant la situation est inédite.

un pays- et pas n'importe lequel -a fait le choix de quitter l'Union européenne. Puissance économique et diplomatique, Londres en était un pilier. Ce constat impose une réflexion sur l'organisation de l'Union européenne elle-même et les réticences qu'elle peut susciter. Je partage ainsi pleinement

Plus qu'un espace de solidarité et d'harmonisation, l'Union européenne est de plus en plus vue comme une machine technocratique et un espace de concurrence déloyale. La France, pourtant aux origines mêmes de la communauté européenne, n'est pas épargnée : « Même atténuée, l'ombre du Frexit demeure », comme le titrait au mois de décembre dernier. La privatisation passée ou à venir de plusieurs entreprises et services publics et la gestion parfois erratique de la crise sanitaire n'ont fait que donner des arguments supplémentaires

En premier lieu, contrairement à ce que souhaitait Boris Johnson, l'Europe n'aura pas, à ses portes, un concurrent britannique non tenu par les normes sanitaires, sociales et environnementales. Cela aurait été une catastrophe à tous les niveaux pour les Européens et leurs entreprises. En second lieu- c'est un nouvel élément à mettre au crédit de Michel Barnier -, les eaux les plus poissonneuses de l'espace européen ne seront pas fermées. Mieux, l'abandon de 60 % des prises des pêcheurs européens a été largement revu à la baisse : il a été fixé à 25 % pour les cinq prochaines années. Cette situation reste toutefois moins favorable aux pêcheurs que la politique commune européenne. Si la Commission européenne commence à rattraper son retard, les délivrances de licences aux pêcheurs ont traîné. Les ports des Hauts-de-France ont fortement pâti de cette situation. Il faut rappeler que 70 % de la pêche artisanale et 96 % de la pêche hauturière de Boulogne-sur-Mer, par exemple, se font dans les eaux britanniques. Or, il y a quinze jours, seuls seize des cent cinquante bateaux avaient obtenu le précieux sésame leur permettant de travailler. À Dunkerque, la pêche artisanale, déjà dramatiquement affaiblie par la concurrence et la diminution des ressources halieutiques causée par la pêche électrique, risque de disparaître totalement. Sur ces deux sujets, et c'est mon premier point d'inquiétude, cet accord n'est que temporaire. La bonne nouvelle est que cela implique un dialogue nourri entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ; la mauvaise est que la situation reste instable et pourrait se dégrader. Ainsi, les Européens ont échoué à mettre en place un mécanisme d'alignement dynamique des normes. Je parlais tout à l'heure des évolutions que devait opérer l'Union européenne pour maintenir l'adhésion volontaire des États membres. La question de la production responsable doit faire partie des chantiers prioritaires et nous pouvons espérer un renforcement des normes dans les années à venir. De fait, l'absence de mécanisme de réalignement risque de conduire à des normes britanniques en deçà des standards européens. Il ne faudrait pas que, d'un côté, l'Union européenne se résigne à ne pas renforcer la protection des Européens et que, de l'autre, on se retrouve dans la situation tant redoutée de pêche, ne risquons-nous pas d'assister, en 2026, à une reprise en main britannique de ses eaux poissonneuses ? La question se pose. L'Union européenne peut-elle garantir la protection des pêcheurs européens, lorsque Londres pourra renégocier annuellement avec, à n'en pas douter, l'ambition d'augmenter le taux d'abandon des prises européennes ? Tout reste à faire dans ce domaine. La City reste une plaque tournante essentielle de la finance mondiale. Les annonces récentes de Boris Johnson doivent nous inquiéter. Il envisage en effet de créer dix ports francs sur son territoire, à l'instar de ceux qui existent au Luxembourg ou en Suisse. Nous pourrions ainsi avoir à nos portes un « Singapour sur Tamise Il y a bien eu quelques transferts en direction d'Amsterdam, de Dublin et même de Paris, mais la suprématie de la City n'est pas entamée sur le fond. Les récentes révélations OpenLux doivent, plus que jamais, appeler l'Union européenne à agir résolument contre les paradis fiscaux en son sein. encore un axe sur lequel l'Union européenne doit impérativement travailler. Comment s'étonner d'un rejet de l'Union européenne quand on assiste, dans le même temps, à une chasse aux services publics à l'échelon européen, à un refus permanent de politiques fiscales ambitieuses et solidaires comme la taxation des transactions financières trop souvent, à une indifférence coupable en ce qui concerne les paradis fiscaux ? Cet accord de coopération constitue, à bien des égards, la conclusion d'un épisode qui marquera l'histoire européenne. Ce dernier doit nous obliger à réinterroger le fonctionnement et la visée de l'Union européenne. C'est d'autant plus central quand on voit avec quelle difficulté le moindre acte de solidarité entre ses pays membres est âprement négocié, à l'image du plan de relance européen. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 24 décembre dernier, un accord de commerce et de coopération a été trouvé de justesse entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il a permis d'éviter un et une sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais certains points de l'accord et leurs effets suscitent toujours inquiétudes et interrogations. Je pense à l'accord conclu sur la pêche ainsi qu'à l'impact du Brexit sur les ports du nord-ouest de la France, particulièrement ceux de Normandie, région dont je suis élue tout comme cinq collègues de mon groupe. Ces ports sont aujourd'hui affaiblis, voire en difficulté économique, en raison de la perte brutale d'activité sans précédent liée à la covid-19. Quasiment toutes les compagnies ferries transmanche annoncent ou mettent en oeuvre des plans sociaux et les exploitants portuaires

Pour toutes ces structures, le départ annoncé du Royaume-Uni de l'Union européenne les a obligées à anticiper la mise en oeuvre de lourds travaux d'aménagement des terminaux pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences en matière de circulation des marchandises et des personnes. Pour les ports normands, la facture s'élève déjà à 8 millions d'euros et elle risque de largement s'alourdir par la nécessité d'installer un poste de contrôle vétérinaire sur le terminal du port d'Ouistreham. Consciente de ces impacts économiques, l'Union européenne a proposé, au mois de décembre dernier, la création d'un fonds d'ajustement au Brexit ayant pour objet de fournir une aide simple et rapide aux secteurs les plus durement touchés par le Brexit. Cette initiative est louable, mais les critères arrêtés pour la répartition de ce fonds entre les États membres posent question. Par exemple, la période de référence pour l'admissibilité des dépenses démarre actuellement au 31 juillet 2020. Or, monsieur le secrétaire d'État, vous imaginez bien que les ports français n'ont pas attendu l'été dernier pour engager de lourdes modifications de leurs infrastructures. Nous espérons que leurs dépenses pourront être éligibles et bénéficier des crédits de ce fonds, et ce rapidement. Cette question est absolument cruciale ! Dans ce contexte, j'appelle votre attention sur le fait que les ports et compagnies devront, en plus, mettre en oeuvre dans quelques mois la directive directive dite, ou système d'entrée et de sortie de l'Union européenne, avec le risque d'un encombrement des terminaux déjà soumis à de fortes tensions. D'ores et déjà, les échanges, notamment en ce qui concerne les produits frais, sont nettement moins fluides. Les installations de l'industrie française de transformation font d'ailleurs état de difficultés significatives. Durant le mois de janvier 2021, les importations de poissons britanniques auraient diminué en volume, mais également en qualité. Si, dans le domaine de la pêche, sujet évoqué par le président de la commission des affaires européennes, l'accord est plutôt satisfaisant, il reste provisoire et n'est que partiellement mis en oeuvre. d'État, pouvez-vous nous éclairer sur les pistes de négociations pour le secteur après le mois de juin 2026 ? Reste le cas des îles anglo-normandes, dont le statut particulier au sein même des zones de pêche britanniques a été remis en cause par l'accord de commerce et de coopération, ayant pour conséquence de fragiliser l'accord de la Granville entre la France et le Royaume-Uni. Les navires français se trouvent désormais dans l'obligation d'obtenir une autorisation pour opérer dans ces eaux. Des licences ont été délivrées sans trop de difficultés sur une base provisoire par les autorités de Guernesey, mais il n'en est pas de même pour le gouvernement de Jersey.

à saluer l'implication sans faille et le travail déterminé depuis 2016. Il aura permis, en dépit des conséquences malheureuses qu'engendre et que continuera, hélas, d'engendrer le Brexit, une sortie par le haut,

nous voilà réunis pour débattre du contenu de l'accord de partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, obtenu à l'arraché le 24 décembre dernier et en application provisoire depuis le 1janvier 2021, en attendant sa ratification par le Parlement européen au mois d'avril prochain, alors dernier. Comme pour toute négociation, cet accord est un compromis, qui permet à l'Union européenne de préserver les principes essentiels du marché unique et d'éviter un dumping sauvage de nos voisins, et qui permet à la Grande-Bretagne de sauver la face tout en renonçant à revoir à la baisse l'ensemble des législations et normes sociales, environnementales et climatiques européennes, contrairement aux annonces initiales du gouvernement Johnson. Les clauses de sauvegarde, clauses miroirs, mesures unilatérales de rééquilibrage et clauses de revoyure sont autant d'outils à la disposition de l'Union européenne pour maintenir une concurrence équitable dans la durée.

la politique étrangère, la sécurité extérieure et la coopération en matière de défense, la politique spatiale, l'enseignement supérieur, les politiques d'asile et d'immigration avec la fin de l'application de l'accord de Dublin, ainsi que l'avenir des services financiers à la suite de la perte de passeport européen. Autant de sujets qui devront faire l'objet de futures négociations. Ensuite, il y a ce qui a été acté, mais qui fait déjà l'objet de remise en cause, en particulier la question nord-irlandaise et le fameux. D'entrée, D'entrée, la mise en oeuvre du protocole s'est heurtée à la réalité, aux difficultés techniques, à l'engorgement des circuits de distribution et a amené les uns et les autres à invoquer l'article 16 du protocole, renforçant ainsi les doutes sur l'applicabilité de celui-ci. D'autres sujets devront retenir notre vigilance comme l'accord provisoire sur la pêche, dont les négociations pluriannuelles risquent de remettre en cause les fragiles équilibres de la politique commune, les inconnues concernant les droits des ressortissants européens résidant au Royaume-Uni, les interrogations pesant sur les appellations d'origine insuffisamment protégées et la protection des données personnelles pour lesquelles le RGPD ne restera applicable que jusqu'au mois de juillet 2021.

il est plus vraisemblable que les États membres, au regard de l'urgence, aient renoncé à demander que soient vérifiées les dispositions qui pourraient relever de la mixité et donc de la ratification par les parlements nationaux. Si l'on peut en comprendre la nécessité politique, il ne faudrait pas, pour autant, que cela crée un précédent juridique et que l'on renonce, pour les futurs accords commerciaux- par exemple l'accord qui s'annonce entre l'Union européenne et la Chine -, à tout droit de regard national.

Le suivi de l'accord sera donc assuré par un conseil de partenariat coprésidé par le commissaire Maroš Šefčovič et le ministre britannique Michael Gove. Ce conseil supervisera la mise en place de multiples comités de pilotage et groupes de travail composés de fonctionnaires qui échapperont à tout contrôle parlementaire. à la vigilance, car ce contrôle ne concerne pas uniquement une mise en oeuvre technique de l'accord, il couvre de réels enjeux politiques. Pour reprendre les mots de l'ancien négociateur en chef Michel Barnier, le Brexit nous aura donc conduits à un accord « perdant-perdant ». Nous devons en tirer toutes les conséquences. Si notre envie d'avancer ensemble à vingt-sept doit rester inébranlable, il est nécessaire de nous interroger sur ce qui a conduit à cette séparation. Il s'agit non pas de se tourner vers le passé, mais d'identifier les failles qui ont conduit nos amis britanniques au Brexit, de sorte d'être capable de désamorcer le sentiment d'éloignement de l'Europe, d'en tirer les leçons pour l'avenir, afin que le projet européen suscite à nouveau l'adhésion de nos concitoyens. Après la création de l'euro, l'Union européenne a fonctionné sur ses acquis. Elle a, pour l'essentiel, accompagné une libéralisation sans frein, une dérégulation tous azimuts, l'abandon des services publics, la montée des inégalités et le risque climatique. Cette posture Cette posture idéologique ne l'a pas prémunie contre une mondialisation exacerbée dont ses citoyens paient le prix, tout comme les territoires de l'Union européenne dont les inégalités de développement opposent de plus en plus villes et territoires ruraux. Le Brexit doit nous servir d'alerte et nous permettre d'envisager une réorientation de l'Union européenne qui réenchante le rêve européen.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis sa création, l'Union européenne poursuit un rapprochement toujours plus fort entre ses peuples et ses membres. Le Brexit va totalement à rebours de l'histoire de la construction européenne. Le départ de l'un de ses membres oblige l'Union européenne à analyser ses faiblesses et ses échecs. La première des faiblesses est la règle de l'unanimité sur certains sujets majeurs. Force est de constater que ce qui fut longtemps un atout est désormais synonyme de prise d'otage, comme l'a mis en lumière le blocage du plan de relance européen

ce ne sont là que quelques exemples. Je salue le travail vertigineux accompli par le négociateur et son équipe pour conclure l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne : ce fut un véritable tour de force jusque dans les derniers instants. à côté de la durée exceptionnellement courte des négociations, les discussions sont, elles aussi, inédites. C'est en effet la première fois que l'Union européenne travaille à l'éloignement plutôt qu'au rapprochement de l'un de ses partenaires. Michel Barnier l'a très bien exprimé lors de sa récente audition, en déclarant que nous avons négocié la divergence réglementaire et non la convergence. C'est pourquoi l'application de l'accord est à mon sens cruciale. Les tensions entre Britanniques et Européens sont palpables et le moindre incident peut prendre des proportions telles que l'équilibre s'en trouvera fragilisé. la mise en oeuvre pour le moins compliquée du protocole concernant l'Irlande du Nord est symptomatique. Nous sommes encore loin d'une relation apaisée et il faudra probablement quelques années et d'autres crises pour parvenir à plus de stabilité. Nous devrons être vigilants pour protéger nos intérêts. Il ne faudra pas faiblir si les règles ne sont pas respectées et si nos peuples sont lésés. En effet, si nous sommes encore dans des règles communes, la divergence réglementaire nous guette. À ce titre, ce titre, les parlements nationaux auront un rôle d'alerte essentiel, tout comme les citoyens. Monsieur le secrétaire d'État, nous sommes prêts à prendre notre part pour la mise en oeuvre stricte de cet accord. Quels sont nos moyens concrets d'action ?

conséquences. Il faudra prêter une attention particulière à l'organisation des liaisons commerciales et des contrôles de produits venant du Royaume-Uni, que ce soit les ports français, belges ou néerlandais. derniers mois, la France a subi plusieurs cyberattaques qui ont touché des collectivités territoriales et des centres hospitaliers. Elles rappellent que la sécurité est essentielle et qu'une coopération dans ce domaine est inévitable. J'espère que le dialogue régulier prévu par l'accord permettra un espace d'échange et d'innovation.

exclus des discussions, pour lesquels il faudra absolument trouver un cadre commun de coopération. Le premier point concerne les frontières et la politique d'asile et d'immigration. Alors que le règlement de Dublin ne s'applique plus au Royaume-Uni, quelles sont les réflexions sur la possibilité d'un accord futur avec l'Union La France et le Royaume-Uni travaillent de concert sur ce sujet depuis longtemps. Monsieur le secrétaire d'État, comment envisagez-vous les prochains mois et des discussions sont-elles prévues sur ces sujets ? Le second point s'articule autour de la politique extérieure, de sécurité et de défense. ait été exclu des négociations, nous allons devoir coopérer. Le contexte international actuel nous oblige à développer une action concrète et commune. L'Union européenne doit regagner en autonomie et les discussions avec le Royaume-Uni ne peuvent pas se faire exclusivement à travers les accords de Lancaster House. soulève, une nouvelle fois, les problématiques de l'Europe de la défense ou d'un volet européen au sein de l'OTAN. Quelles sont les pistes de réflexion du côté tant français qu'européen ? Après avoir travaillé à la sortie des Britanniques de l'Union européenne, nous devons nous concentrer sur nous, Européens. Michel Barnier l'a très justement souligné, il faut se rendre compte de la valeur ajoutée de l'Europe. Nous devons continuer à créer cette valeur ajoutée : de nombreux sujets réclament notre attention et notre coopération. Le rêve européen se poursuit, mais il est gravement menacé. Le Brexit nous donne l'occasion de nous interroger sur nous-mêmes et sur la logique européenne. Comme l'écrivait Jean Monnet, « ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste, mais d'être déterminé

Fernique. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en 2016, nous subissions deux coups durs qui obscurcissaient notre horizon : l'avènement de Donald Trump aux États-Unis et le choix du Brexit par une majorité de Britanniques. Ces deux événements successifs ont été lourds de conséquences : le repli, le désengagement des valeurs communes et le rejet des responsabilités solidaires avaient pris la main. Aujourd'hui, l'horizon se dégage quelque peu : les États-Unis engagent une nouvelle trajectoire et la mise en oeuvre du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne s'engage de façon ordonnée.

Le Brexit provoquera de considérables changements sans effacer pour autant les logiques de l'histoire et de la géographie : l'Union européenne et le Royaume-Uni entretiendront toujours une relation privilégiée et les chances de coopération ne sont pas liquidées. Sur une planète où l'interdépendance est de rigueur, le moyen pour les démocraties de prendre la main est de coopérer. C'est donc, en ce sens, une une évolution encourageante qu'après le temps des outrances et des propos à l'emporte-pièce le gouvernement britannique ait admis qu'un accord avec son très proche et très grand voisin

des dégâts collatéraux : c'est à l'usage que cet accord fera ou non ses preuves. D'ores et déjà, les préoccupations sont sérieuses et nécessiteront une vigilance solide de l'Union européenne qui, jusqu'à présent, n'en avait guère fait preuve dans la gestion de ses accords commerciaux largement marqués par l'ultralibéralisme.

Il serait en effet tentant de mettre le tampon « origine britannique » sur des assemblages de pièces importées produites dans des conditions sociales et environnementales inacceptables pour pouvoir ensuite les répandre dans le marché unique et détruire ainsi nos emplois. l'encadrement sera robuste, nous dit-on, pour empêcher des distorsions de concurrence provoquées par des aides d'État ou par des divergences réglementaires qui régresseraient par rapport au niveau de 2020. On le sait, l'enfer est dans les détails et il est toujours pavé de bonnes intentions. Tout dépendra de la gouvernance et de sa réactivité : notre exigence est forte dans ce domaine. Chacun sait combien nos normes environnementales sont appelées à progresser pour tenir nos engagements. La clause de non-régression ne suffira pas à éviter les divergences dommageables. Il faudra faire preuve d'une grande rigueur. Les instruments sont dans le texte. Tout dépendra de la manière dont la Commission européenne les mettra en oeuvre. Il faudra que le Parlement ait la possibilité effective de réagir s'il se trouvait que l'on reste l'arme au pied. La faiblesse des mesures contre le blanchiment d'argent et contre l'évasion fiscale pose problème. Sur cette dernière, l'accord se borne aux règles de l'OCDE et non à celles de l'Union européenne, qui sont plus strictes. L'accord ne prévoit aucune disposition à l'encontre du réseau britannique de zones offshore, qui représente tout de même plus du tiers des dommages causés par les paradis fiscaux à l'échelon mondial- excusez du peu ! L'Union européenne elle-même a encore le ménage à faire en son sein. L'accès des services financiers britanniques au marché unique n'est pas pour demain. S'il devait en être question à l'avenir, il devrait être conditionné à des engagements sans ambiguïté de la part de Londres en faveur de la lutte contre l'évasion fiscale et de la transparence financière. Au moment où la pandémie creuse nos déficits publics, il serait irresponsable de laisser faire ces pratiques fiscales et, pour reprendre les mots d'Éric Bocquet, de laisser s'instaurer un « Singapour sur Tamise » à nos portes. Sur la protection des données, nos inquiétudes sont très sérieuses, puisque, au-delà du 1 juillet prochain, le cadre n'est pas fixé. Il serait inacceptable que le Royaume-Uni puisse maintenir les flux de données avec l'Union européenne, alors qu'il s'éloignerait considérablement du modèle européen de protection des données basé sur les droits. le débat sur cet accord nous amène plus globalement à considérer les motivations populaires qui ont amené à cette volonté britannique de divorce. Les mécanismes sont toujours à l'oeuvre au sein de l'Union européenne désindustrialisation, relégation sociale, délitement des biens communs et des services publics, crise démocratique ... Autant de béances qu'il faut réparer. Je conclurai sur les mots d'une petite fille, Stella, qui, du haut de ses 10 ans, m'a lâché dimanche, en jetant un coup d'oeil sur mon écran Le Brexit, c'est tout pourri : si on continue comme cela, on se retrouvera chacun tout seul. » À elle et à tous les autres, notre Europe doit faire comprendre que l'on ne continuera pas ainsi !

au centre du monde et passant des accords de libre-échange bilatéraux avec un ensemble d'autres pays ou d'autres régions- les États-Unis, les pays du Commonwealth et l'Asie.

très prudente et n'a accordé que très peu d'équivalences financières, ces certificats qui permettent à une institution britannique d'exercer et

que le Royaume-Uni voudra bien accepter. La France doit jouer un rôle

Dans quelques semaines, un premier bilan de l'accord entré en vigueur le 1 janvier de cette année sera dressé. Quoi de plus naturel ? Évidemment, chacun a conscience des effets de la crise sanitaire, dont la gravité et la durée masquent les perspectives.

que souligner : celle des questions de défense, comme l'a souligné Christian Cambon, son président. Si je regrette, ô combien, le départ de l'Union européenne de nos amis britanniques avec fracas et non sans tourments, je me rappelle que d'autres l'ont fait sans bruit, sur la pointe des pieds, sur les plaines enneigées et glacées du Groenland, en 1982. Vous auriez raison de me dire que comparaison n'est pas raison. La France et le Royaume-Uni sont deux puissances nucléaires, ont un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et représentent 60 % des dépenses européennes de défense et 80 % des dépenses de recherche et développement dans ce secteur.

face à ses demandes, n'a pas jugé « urgent » d'inclure le volet relatif à la défense dans les discussions. C'est somme toute regrettable et loin d'être sans conséquence sur cet épineux sujet, objet de longues et complexes discussions discussions entre la France, l'Allemagne et les vingt-cinq autres pays de l'Union européenne. Faut-il convoquer les discours qui ont accompagné naguère l'impérieuse nécessité de construire l'Europe de la paix ? Doit-on se remémorer l'intelligence collective qu'il a fallu déployer pour la reconstruction de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Aujourd'hui, le rêve d'une défense européenne- je n'ose utiliser le mot « armée » -reste une chimère et laissons de côté la brigade franco-allemande, à laquelle il faudra bien un jour donner corps. Or il apparaît clairement

et que l'on ne soutienne pas que le départ des Britanniques ne change rien, puisqu'ils refusaient de concourir pleinement à la politique de sécurité et de défense commune, alors même qu'ils l'avaient relancée par la déclaration franco-britannique de Saint-Malo de 1998. L'OTAN a été sérieusement affectée par les errements de la présidence Trump et son successeur a bien des chantiers à entreprendre pour que nous puissions espérer un retour rapide à la normale. Or, dans ce monde où les dangers se multiplient, à l'heure où les crises régionales prospèrent et menacent les équilibres élaborés au lendemain de la chute du mur de Berlin,

Elle n'a pas à se préoccuper uniquement des droits des consommateurs et de la libre concurrence. Elle a aussi une citoyenneté à bâtir et à défendre. Pour cela, cela, s'il est indispensable d'analyser le départ du Royaume-Uni, nous devons travailler rapidement, sérieusement, concrètement à l'élaboration de cette défense européenne. Ce chantier n'est pas seulement nécessaire : il est incontournable à l'heure où le multilatéralisme

Il nous faut désormais faire avec, en respectant leur volonté, mais en conservant à l'esprit la nécessité d'une coopération dans de nombreux domaines avec nos voisins d'outre-Manche. Je rappelle la position unique du Royaume-Uni par sa proximité géographique et ses volumes d'échanges avec l'Union européenne. Certes, nous avons vécu les derniers mois de 2020 au rythme des aléas, des doutes et des postures dans les négociations en vue d'obtenir un accord. Le, c'est-à-dire le scénario du pire, a été évité de justesse, mais rien ne sera plus comme avant. De profonds changements sont en cours, qui affectent les citoyens, les entreprises, les administrations publiques et de nombreux acteurs, aussi bien dans l'Union européenne qu'au Royaume-Uni. Ce ne sera plus, comme le souligne le négociateur Michel Barnier. chaque côté du, chacun se rassure et personne ne veut perdre la face, même si, pour le Royaume-Uni, les compromis au cours des négociations n'ont jamais conduit à déroger à l'objectif de restauration de la souveraineté nationale, objectif central de la sortie de l'Union Pourtant, je le crois, le Brexit est une situation perdant-perdant. Il affaiblit l'Europe à l'heure où les États-Unis sont fragilisés et où d'autres puissances décomplexées émergent et s'entendent. Je pense notamment aux rapprochements russo-chinois ou russo-turc. Dans ce contexte, il nous faut poursuivre de manière organisée, comme le prévoit le présent accord, sur de nombreux sujets. Toutefois, des craintes demeurent, notamment liées à l'altération de la confiance au cours des négociations et aux aléas des premières heures d'application. Nous avons pu, avec quelques collègues du groupe de suivi de la nouvelle relation euro-britannique, constater les difficultés et les lourdeurs lors d'une visite à Calais et à Boulogne-sur-Mer. Jusqu'au dernier moment, la question du droit de pêcher dans les eaux du Royaume-Uni a été un obstacle à la conclusion de l'accord.

ont d'abord été ressenties comme un soulagement, elles suscitent des inquiétudes de la part des pêcheurs français et de toute la filière, déjà affectée par la crise du covid.

lorsque l'accord devra être renégocié ? Les pêcheurs britanniques, qui se sont sentis floués, ne désarment pas sur les questions de souveraineté et se plaignent des prises perdues ou gâchées en raison des nouvelles contraintes administratives. Comme l'a signalé Jean-François Rapin, la question des licences persiste. Cette question de l'horizon est cruciale pour la profession, car le coût considérable d'acquisition d'un bateau de pêche implique une longue durée d'amortissement. Dès lors, quel jeune voudra se former et s'engager dans le métier ? Quel banquier voudra lui accorder des crédits importants ? La reconversion, même subventionnée, n'est pas souhaitable. En effet, on sait que la souveraineté alimentaire est l'un des défis du siècle, ce qui fait basculer le sujet de l'économie locale à la préoccupation stratégique. Quel sera l'avenir des ports français dans ce contexte post-Brexit et dans celui d'une économie maritime globale qui continuera d'exploser ? La volonté affichée de faire de la France le « hub de l'Europe » nécessitera beaucoup d'efforts. Les ports d'Anvers et de Rotterdam, déjà leaders, sortiront-ils renforcés à notre détriment ? Les ports sont des actifs stratégiques. Les Chinois, avant nous, l'ont bien compris, eux qui investissent partout dans le monde et prennent progressivement le contrôle des opérateurs portuaires et du transport de conteneurs. Je note avec intérêt la coopération étroite prévue par l'accord entre les autorités policières et judiciaires nationales et l'échange rapide de données essentielles. Cela permettra, en outre, une coopération efficace entre le Royaume-Uni, Europol et Eurojust. La criminalité internationale, le terrorisme et la cybercriminalité sont, hélas, des secteurs en croissance, qui menacent nos sociétés. Face à ces dangers, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent rester des priorités. Enfin, si les questions de défense ne figurent pas dans le présent accord, elles représentent un autre volet de la nécessaire coopération avec les Britanniques, étrangères l'a à juste titre parfaitement rappelé. Nous devons poursuivre dans l'esprit des accords de Lancaster House, qui ont fêté leurs dix ans récemment. Les enjeux opérationnels et industriels sont importants. En conclusion, nous avons de nombreux points de convergence et des intérêts communs avec les Britanniques. Le bon sens nous commande de poursuivre dans cette voie coopérative, mais les relations privilégiées avec les États-Unis et le Commonwealth assurent déjà à ces derniers une grande ouverture sur le monde. De plus, le Royaume-Uni entend bien revenir « au-delà de Suez » par sa demande d'adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique, pour se rapprocher des économies asiatiques en forte croissance, et son récent accord de libre-échange avec le Japon. Son intérêt stratégique pour l'Indopacifique se confirme, de même que sa présence militaire, grâce à des capacités augmentées de projection de puissance. Dès lors, compte tenu de la marche du monde, y aura-t-il une véritable volonté de la part des Britanniques d'investir durablement dans la relation avec l'Union européenne

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 24 décembre dernier, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord de commerce et de coopération. Le groupe Union Centriste s'en réjouit. Cet accord vient compléter l'accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Nous saluons les efforts du Gouvernement pour protéger nos intérêts je vous remercie de la fermeté dont vous avez fait preuve sur le sujet à chacune de vos interventions. Je souhaite également souligner la qualité de l'action de Michel Barnier. Son sens du collectif a permis aux Vingt-Sept de rester soudés de bout en bout de la négociation. Face aux tergiversations des Britanniques, qui ont toujours peiné à fixer l'objectif à atteindre, Michel Barnier a souvent répété : « L'horloge tourne ! » En effet, ce sont les Britanniques qui nous ont imposé le 31 décembre 2020 comme date butoir pour la négociation d'un accord. Boris Johnson a annoncé la conclusion d'un traité à la veille de Noël et n'a laissé que trois jours ouvrables avant la date de son entrée en vigueur. Les entrepreneurs ne remercient pas le Premier ministre britannique. Premier ministre britannique. « Personne ne sait comment faire et nous découvrons des problèmes partout ! », m'a confié hier un expert-comptable britannique qui s'occupe de dizaines de PME. À titre d'exemple, nous avons vu apparaître, côté britannique, des frais de douane applicables aux envois dont la valeur dépasse 130 livres sterling. De nombreuses entreprises n'ont pas anticipé de se retrouver devant une telle lourdeur des démarches relatives à la TVA. Ainsi, certaines ont payé la TVA à deux reprises. Elles m'ont dit avoir cessé de commander en ligne pour se fournir depuis l'Union européenne, car elles ne maîtrisent plus leurs coûts d'approvisionnement. Comment le Gouvernement prévoit-il de mesurer l'impact de l'accord sur les PME françaises ? avez-vous prévu des mesures d'accompagnement spécifiques afin de leur éviter une perte de compétitivité outre-Manche ? Autre difficulté, nos entreprises établies en Grande-Bretagne ne peuvent plus accueillir de jeunes étudiants stagiaires venant de France.

Les services financiers ne font pas partie de l'accord alors que l'industrie des services financiers pèse très lourd : elle représente 7 % du PIB britannique. Les entreprises britanniques du secteur ont délocalisé au moins 7 500 emplois du Royaume-Uni vers Paris, Francfort, Dublin ou Amsterdam. Comment les places financières européennes comptent-elles pérenniser les avantages acquis grâce à la migration des activités d'de certaines grandes banques internationales ? Comment peuvent-elles fidéliser ces hauts cadres dirigeants fortement touchés par la fiscalité européenne ? Dans ce secteur dématérialisé qu'est la finance, le Brexit fait d'autant plus peur qu'il semble une opportunité de s'affranchir des règles européennes. Comment éviter que la rupture de cadre et d'équivalence entre Londres et l'Europe ne donne lieu à une concurrence déloyale ? Les grands groupes financiers ont mis leurs oeufs dans différents paniers et implanté leurs activités dans différents pays européens, notamment par crainte de voir un autre pays sortir à son tour de l'Union européenne. Comment leur donner confiance en la solidité et la pérennité de l'Union européenne ? Nous ne sommes pas au bout du chemin. L'accord de commerce et de coopération laisse de nombreux points sectoriels à négocier. Certains observent que les relations commerciales après le Brexit sont comme un oignon : chaque fois que vous enlevez une couche, vous en découvrez une autre, qui vous fait pleurer un peu plus. La combinaison Brexit-covid rend la situation très difficile à supporter pour ceux qui vivent à cheval entre les deux pays. À quelle date le Royaume-Uni et la France prévoient-ils de supprimer la raison impérieuse pour pouvoir passer d'un pays à l'autre ? Bravo ! La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon court propos sera consacré aux conséquences du Brexit sur la défense européenne, sur la problématique irlandaise ainsi que sur les règles relatives au regroupement familial des demandeurs d'asile.

Aujourd'hui, les dispositifs existent et la question de l'ambition de l'Europe ne tient pas tant à l'argent qu'elle attribuera au Fonds qu'à la vision de ce que doit être son autonomie stratégique, à l'heure où la puissance américaine a fait d'elle un théâtre périphérique. Le contexte récent a permis de clarifier plusieurs points, et non des moindres. Les années Trump auront eu le mérite d'obliger l'Union européenne à mesurer l'impérieuse nécessité d'exister sur les terrains pourtant privilégiés de la souveraineté nationale : la défense et la politique étrangère. La crise sanitaire a tristement ouvert les yeux des Vingt-Sept quant à la nécessité d'une plus grande indépendance dans des domaines clés, comme la santé ou encore les technologies de l'avenir. au Brexit, il a privé les Vingt-Sept du paravent britannique bien utile pour cacher leurs divisions et leurs degrés d'ambition variables sur les questions de défense.

que, avec la France comme seul acteur majeur depuis le Brexit, la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne pouvait être relancée, voire renouvelée l'Irlande. L'épisode avorté d'un retour des contrôles à la frontière irlandaise pour surveiller les exportations de vaccins en dehors de l'Union européenne a agi comme un révélateur. Michel Barnier l'a déclaré et nous sommes nombreux à partager ce constat : « L'activation de la clause article 16 était une erreur. » N'était-ce qu'une erreur de méthode ? Le problème est bien plus profond. L'accord de retrait négocié en 2019 et dans lequel a été organisée la question de la frontière irlandaise préconisait une relation future plus étroite que ce que prévoit l'accord commercial signé au mois de décembre 2020. Monsieur le secrétaire d'État, s'il nous faut trouver des solutions pour limiter les impacts du Brexit sur le processus de paix en Irlande, il nous faut surtout maintenir un front commun européen, une union qui nous permettra de faire face à la longue série d'épisodes à venir. Ne nous y trompons pas : il y en aura au regroupement familial des demandeurs d'asile. Depuis le 1 janvier 2021, les seules options qui s'offrent aux demandeurs d'asile pour rejoindre le Royaume-Uni depuis la France, quels que soient leur âge, leur vulnérabilité ou leurs attaches outre-Manche, sont des voies irrégulières et dangereuses, tout particulièrement pour les enfants. En effet, les dispositions du règlement communautaire dit Dublin III ont cessé de s'appliquer. Il s'agissait pourtant d'un dispositif légal et reconnu combattre les passeurs et les filières de criminalité organisée. Deux mois après le Brexit et la publication de la déclaration conjointe sur l'asile, nous ne disposons d'aucune précision quant à l'agenda ou au cadre dans lequel des discussions seront engagées.

et agissent au plus vite pour mettre en place un nouveau mécanisme garantissant le droit à la réunification familiale. À défaut, pouvons que redouter encore davantage de tragédies sur le littoral français. Le grand Calaisis en sait quelque chose ... Mes chers collègues, depuis 2018, les traversées sur des embarcations de fortune ont été multipliées par dix. Vous l'aurez compris, la mobilisation des autorités est vitale et essentielle, associée à la plus grande vigilance sur l'efficacité de l'accord en question. La parole est à M. Alain Cadec. Madame

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est le résultat d'un processus long et pénible de plus de quatre ans. Il convient de féliciter Michel Barnier de l'excellent travail réalisé, d'abord pour ce qui concerne l'accord de sortie, et ensuite pour ce qui concerne l'accord de commerce et de coopération. Cependant, on peut difficilement parler de « succès » : comme Michel Barnier l'a souvent souligné, il s'agit d'un scénario « perdant-perdant » dans lequel tant l'Union européenne à vingt-sept que le Royaume-Uni se retrouvent dans une situation dégradée par rapport au Sur le Sur le plan commercial, un accord de libre-échange n'est pas une union douanière et la circulation des marchandises, même en exonération de droits de douane, est beaucoup moins fluide, notamment en raison des règles d'origine, des formalités douanières et du contrôle du respect des normes sanitaires et phytosanitaires. Les opérateurs commerciaux des deux côtés s'en sont déjà rendu compte et les choses ne sont malheureusement pas appelées à s'améliorer. Sur le plan politique, les deux parties ressortent affaiblies de l'exercice : le Royaume-Uni perd toute une série d'avantages liés à sa participation aux politiques et programmes de l'Union, ainsi qu'à tout le réseau des accords internationaux conclus par l'Union au fil des années ; et l'Union européenne, quant à elle, « pèse moins lourd » à vingt-sept qu'à vingt-huit et se retrouve flanquée d'un nouveau concurrent et d'un partenaire difficile à ses portes. La négociation de l'accord bilatéral de commerce et de coopération a donc essentiellement consisté en un exercice de limitation des dégâts. Il n'a pas été facile et, à plusieurs reprises, les deux parties se sont fait peur en voyant approcher la terrifiante possibilité d'une « chute de la falaise »- , c'est-à-dire c'est-à-dire d'un. L'accord obtenu est un accord d'association assez classique, lequel, à certains égards, va même moins loin, en termes de coopération, que certains accords avec d'autres partenaires de l'Union. Il est néanmoins sans précédent sur le plan commercial par le fait qu'il permet des échanges de marchandises sans aucun droit de douane ni quota, sans la moindre exception ou période transitoire, pour l'agriculture et la pêche, par exemple. Je me réjouis que l'Union européenne ait imposé un cadre juridique et institutionnel unique pour la gestion de tous les volets de la relation bilatérale. Le précédent suisse, notamment, a démontré combien l'option d'une série d'accords bilatéraux plus ou moins bien reliés les uns aux autres est problématique, à la fois sur le plan technique et sur le plan politique. Le « saucissonnage » aurait été dramatique pour l'Union européenne. La question délicate de la circulation des personnes était déjà réglée par l'accord de retrait en ce qui concerne les droits acquis des citoyens britanniques dans l'Union européenne et ceux des citoyens européens au Royaume-Uni. Dans le futur, l'accès des citoyens européens au territoire et au marché du travail britanniques sera plus difficile que par le passé- c'était sans doute l'un des principaux objectifs du Brexit -, mais des garanties minimales réciproques ont été obtenues en matière de visas et de protection sociale. La participation du Royaume-Uni à certains programmes européens reste possible si les deux parties le souhaitent et à des conditions appropriées pour un pays tiers, notamment en termes de participation financière. La sortie du Royaume-Uni du programme Erasmus+, pour des raisons essentiellement politiques, est cependant une énorme déception pour tous les jeunes potentiellement concernés de part et d'autre. Une autre grande déception concerne les garanties d'une concurrence loyale, ce qu'il est convenu d'appeler le, qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous aurions pu espérer. La négociation a mis en évidence l'intention du Royaume-Uni de concurrencer l'Union en activant tous les leviers à sa disposition et en tirant pleinement parti de sa souveraineté recouvrée en matière réglementaire. L'Union devra donc rester vigilante et ne pas hésiter à protéger ses intérêts.

en raison non seulement de l'importance des intérêts économiques en jeu, mais aussi de sa charge symbolique et politique particulièrement élevée. L'équation à résoudre était très complexe. Le compromis trouvé est forcément source de frustration pour nos pêcheurs puisque, comme dans d'autres domaines, il représente une dégradation sensible par rapport au. On On peut néanmoins considérer que le résultat aurait pu être bien pire, puisque le transfert de quotas au profit du Royaume-Uni ne concernera finalement que 25 % des possibilités actuelles sur cinq ans au lieu des 80 % réclamés initialement par Boris Johnson. Il faudra surtout bien veiller à préserver nos possibilités d'accès aux eaux britanniques, qui ne seront plus garanties au-delà du 30 juin 2026,

Ce protocole n'est pas le résultat de la négociation qui vient de s'achever : il a été conçu dans le cadre de la négociation précédente sur l'accord de retrait. Le problème de sa mise en oeuvre effective ne se pose cependant que depuis le 1 janvier dernier, alors que le Royaume-Uni est désormais sorti de l'union douanière et du marché unique. Pour éviter le rétablissement d'une frontière visible entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, le protocole a mis en place des dispositions extrêmement complexes qui, pour l'essentiel, maintiennent le territoire d'Irlande du Nord dans l'union douanière et le marché unique, imposent des contrôles stricts sur les échanges entre ce territoire et le reste du monde, y compris la Grande-Bretagne, et s'en remettent aux autorités douanières britanniques présentes en Irlande du Nord pour les exercer. Ce système n'est pas dénué de failles intrinsèques. L'une d'entre elles s'est déjà révélée de manière spectaculaire au sujet des contrôles que l'Union européenne a récemment voulu instaurer sur les exportations de vaccins. Pire encore, son efficacité dépend entièrement de la bonne coopération d'autorités britanniques, qui ont fait preuve jusqu'ici d'une extrême mauvaise volonté. Je crains donc que l'intégrité de l'union douanière et du marché unique, qui était l'un des grands objectifs des négociations, ne soit pas assurée à travers cette véritable « usine à gaz » du protocole sur l'Irlande. Je prévois malheureusement de sérieux dysfonctionnements dans les mois qui viennent avec le risque de répercussions importantes sur la situation politique en Irlande-

Madame la présidente, monsieur le président Christian Cambon, monsieur le président Jean-François Rapin, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux d'avoir l'occasion de répondre

Europe. Les accords du Vendredi saint sont fondés dans un enracinement européen : c'est grâce au marché intérieur et aux règles européennes que cette dissociation entre deux entités politiques et une entité économique avait été rendue possible, voilà un peu plus de vingt ans. N'oublions pas le rôle qu'avait joué notre cadre européen dans cet accord de paix.

Je veux être précis sur les développements récents, puisque nous allons vivre durablement avec ce protocole et ces complexités. Les frictions que nous constatons parfois dans le commerce

dont nous devons tirer des conséquences, en essayant de les minimiser pour l'Irlande et pour l'Union européenne, mais dont nous ne pouvons faire fi, comme si le Royaume-Uni était resté dans le marché unique, dans l'union douanière et dans l'Union européenne. Nous ne devons pas nous tromper quant aux responsabilités à cet égard. Nous ne devons pas être dupes de

aux Britanniques de l'appliquer intégralement ; et c'est l'application intégrale de l'accord qui peut permettre une discussion pragmatique sur d'éventuelles flexibilités, notamment pour les périodes de grâce. Nous ne devons pas inverser l'ordre des paramètres. À l'instant où nous parlons, nous apprenons que le Royaume-Uni a

C'est évidemment illégal et inacceptable. C'est seulement dans le cadre d'une discussion, lorsque le respect du protocole aura été préalablement garanti, que nous pourrons envisager des flexibilités, mais certainement pas de manière unilatérale. Je tenais à le rappeler à cette tribune. Très bien ! En En ce qui concerne la négociation, nous avons ensuite essayé de forger le cadre d'une relation future avec le Royaume-Uni : ce fut

alimentaires, sanitaires ... Toute divergence réglementaire jugée significative peut donner lieu, de part et d'autre, à des mesures de compensation

reste lié à la France, à l'Union européenne et à l'Europe par des liens humains, affectifs, culturels et par des valeurs communes que nous partagerons encore. Il était important de ne pas se tourner le dos à l'issue de cette période de négociations difficiles.

par les opérateurs économiques, lesquels pourraient ainsi signaler toute difficulté, tout écart, toute divergence dans l'application de cet accord et le respect des normes.

de concurrence, peut servir de modèle à une réforme de la politique commerciale européenne à l'égard d'autres partenaires. Nous connaissons les débats sur le respect des normes environnementales et sociales, en particulier, que nous avons légitimement avec d'autres partenaires commerciaux plus éloignés géographiquement. La politique commerciale européenne mérite d'être réformée en s'inspirant de cet accord.

elle a aussi laissé un certain nombre de traces dans nos relations. Nous avons perdu des habitudes de travail en commun que nous devons retrouver. Je ne pense pas que nous les ayons perdues en matière de sécurité et de défense, notamment en matière opérationnelle, mais nous devons sécuriser cette relation, un peu plus de dix ans après les accords de Lancaster House et préparer un sommet bilatéral pour évoquer cette coopération dans les prochains mois. Il faudra aussi définir un cadre de coopération, non pas seulement franco-britannique, mais euro-britannique, qui n'existe pas aujourd'hui. Ce sont les Britanniques qui n'ont pas souhaité intégrer cette dimension dans l'accord. Regrettons-le, mais travaillons sur la suite. La France a fait un certain nombre de propositions,

Quelques jours avant la conclusion de l'accord sur la relation future, les ministres de l'intérieur français et britannique ont signé un nouvel accord de coopération avec un renforcement des financements britanniques

d'asile, notamment celle du retour, puisque nous ne sommes plus dans le cadre du règlement de Dublin, nous avons le choix entre la voie d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et celle d'un accord bilatéral. Il me semble que la plus pragmatique serait celle d'un accord bilatéral spécifique pour

probablement d'autres coopérations en matière académique, scientifique ou étudiante à l'avenir. C'est notre intérêt commun. À court terme, nous devons renforcer notre programme Erasmus, notre programme Horizon Europe en matière de recherche dans l'Union européenne, avec des pays tiers qui cherchent à s'y associer. C'est ainsi que nous faciliterons la mobilité de nos étudiants et le financement de notre recherche. Vous l'avez souligné par différentes formules,

Nous avons démontré, dans cette négociation, notre capacité à défendre notre unité- peut-être au-delà de ce que nous espérions -, notre capacité à imaginer. Je suis convaincu que le plan de relance européen,

Nous avons consolidé notre unité et témoigné de notre force. Nous devons maintenant démontrer notre agilité face au Brexit et à ce que d'éminents responsables politiques auraient appelé, en d'autres temps, des « expérimentations hasardeuses

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

le maintien d'une certaine exigence en matière de normes environnementales, sociales et fiscales impose, en toute logique, une augmentation des contrôles aux frontières. Bonne nouvelle, les embouteillages craints du côté français semblent avoir été anticipés intelligemment. Entre le recrutement de 700 fonctionnaires, les 40 millions d'euros investis par les opérateurs transmanche et les aménagements des ports, notamment dans mon département, à Dunkerque, la fluidité du trafic semble être assurée.

régime ? Mauvaise nouvelle, le passage entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord bloque. La zone prend une nouvelle dimension. Ainsi, Dunkerque vient d'inaugurer une nouvelle ligne réservée aux poids lourds et reliant directement Dunkerque à Rosslare. Mais cela conduit aussi à une augmentation du trafic entre les deux Irlande. Les conséquences s'en font déjà ressentir, puisqu'on note de nombreuses pénuries dans les supermarchés nord-irlandais. De plus, à compter du 1 avril, chaque transport de produits alimentaires nécessitera un certificat sanitaire. Étant donné l'intensité des relations commerciales entre les deux territoires, on risque de se retrouver avec des blocages. C'est d'autant plus problématique que, à l'intérieur d'un même camion, on peut trouver 300 à 400 produits alimentaires, ce qui nécessiterait autant de certificats sanitaires différents. Monsieur le secrétaire d'État, l'Union européenne a rejeté le délai demandé par Londres pour normaliser le transit nord-irlandais. Malheureusement, ce sont bien les Nord-Irlandais et les Nord-Irlandaises qui payent le tribut de l'intransigeance de Bruxelles et de Londres.

la sénatrice Morin-Desailly sur la situation de Brittany Ferries. La ligne Rosslare-Dunkerque est un bon exemple d'une opportunité économique nouvelle qui se développe entre l'Irlande et la France. Cela ne compensera pas toutes les difficultés que connaissent, au-delà de la question du Brexit et

est à M. Yves Détraigne. Monsieur le secrétaire d'État, après la prochaine année scolaire, les jeunes Européens ne pourront plus étudier au Royaume-Uni grâce à Erasmus. Les étudiants britanniques ne pourront donc plus obtenir de bourses de l'Union européenne pour étudier sur le continent, et les étudiants européens ne pourront plus accéder aux aux établissements britanniques grâce à un financement de l'Union européenne. Les Britanniques ont en effet considéré qu'ils perdaient trop d'argent avec ce programme, car ils accueillaient plus d'étudiants européens qu'ils n'envoyaient de jeunes Britanniques sur le continent. Pourtant, en rapportant ces dépenses à la participation du Royaume-Uni pour financer Erasmus, le pays engrangeait un bénéfice net, les étudiants étrangers consommant sur place et contribuant à la vie économique du pays. Boris Johnson a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un programme propre au Royaume-Uni, intitulé Alan Turing, pour permettre aux étudiants britanniques d'accéder aux universités européennes, mais aussi aux meilleures universités du monde. À l'inverse, les étudiants européens devront s'acquitter de frais de scolarité aussi élevés que les autres étudiants étrangers - plus de 10 000 euros l'année pour venir étudier au Royaume-Uni. Depuis trente-trois ans, ce pays s'était imposé comme l'un des principaux pays d'accueil des étudiants européens au sein d'Erasmus. C'est donc une décision qui aura des conséquences non négligeables sur les mobilités des étudiants européens, plus particulièrement s'ils sont issus de milieux défavorisés.

M. Gilbert Roger. Monsieur le secrétaire d'État, l'accord prévoit un système de coopération ouvert fondé sur un dialogue régulier, afin d'échanger des informations sur les évolutions des politiques liées au cyberespace, de l'internet, la cybersécurité et la cyberdéfense. Des mécanismes de coopération avec les pays tiers sont prévus, mais ce type de procédure est contraignant et entraîne souvent des délais supplémentaires. Monsieur le secrétaire d'État, pensez-vous que cette coopération, fondée sur le volontariat, permettra de répondre au mieux aux enjeux stratégiques de cybersécurité ? Quel dispositif est prévu pour le signalement des incidents de sécurité, alors que la directive NIS- , qui établit un niveau commun de protection des données, ne prévoit pas de coopération renforcée avec les pays tiers ? Le Royaume-Uni risque-t-il d'être confronté à des difficultés en matière d'enquête sur des actes de cybercriminalité ? de la participation britannique aux exercices en Europe ? Ne craignez-vous pas une coopération moins performante en matière de lutte contre la cybercriminalité ? Enfin, le Brexit

ma question concerne les difficultés des pêcheurs de la côte ouest du département de la Manche, depuis l'abrogation, à la surprise générale, du traité de la baie de Granville, à la suite des accords du Brexit. Signé en juillet 2000, ce traité entre la France et le Royaume-Uni réglementait la pêche à proximité de Jersey et faisait de ce secteur transfrontalier une entité juridique unique permettant de se partager la mer entre voisins. De moins en moins nombreux, les bateaux français sont soumis à des réglementations restrictives : leur accès est encadré par des conditions de licence, de matériel et de quotas. La proximité géographique entre Jersey et les côtes normandes est un cas unique et non délocalisable. Les bateaux qui pêchent dans les trois à douze milles forment une flotte composée de petites unités qui ne peuvent pêcher plus au large. L'accès à cette zone leur est donc indispensable. Dès le mois de janvier, des inquiétudes ont vu le jour et il a été décidé d'une période de cent vingt jours, jusqu'au 30 avril, pour trouver un accord. Cependant, plusieurs incidents ont émaillé les relations avec Jersey. Les licences données jusqu'alors par le comité de pêche sont désormais délivrées par Jersey aux bateaux pouvant justifier d'un nombre de dix jours de pêche. Sur 340 bateaux recensés, 57 ont obtenu leur licence. Les autres ne disposent que de licences provisoires expirant au 1 mai nouveau revirement de la Commission européenne, la débarque de bulots pêchés par des bateaux jersiais est interdite pour un pays tiers, car ces coquillages sont prélevés dans des eaux classées en B. Alors que les pêcheurs normands pêchent ces produits dans les mêmes eaux et débarquent sans problème, les bateaux de Jersey sont refoulés vers Ouistreham ou Saint-Malo, causant un préjudice économique aux ports de Granville et de Carteret. Comme vous pouvez le constater, monsieur le secrétaire d'État, cette situation n'est pas tenable et nos pêcheurs ne doivent pas être les grands sacrifiés sur l'autel de l'accord du Brexit. Qu'entendez-vous faire pour remédier à cette profonde injustice, qui pourrait déboucher sur une situation sociale et économique explosive ?

importantes : il convient d'obtenir, à court terme, les licences les plus complètes ou les plus nombreuses possible. Pour la zone économique exclusive, nous les avons obtenues jusqu'au 30 avril. Pour les îles anglo-normandes, nous les avons également obtenues jusqu'au 30 avril. Nous devons encore les obtenir, obtenir, et ce le plus vite possible, pour la bande des six à douze milles, qui concerne avant tout les Hauts-de-France. Au-delà du 30 avril, c'est le point que vous souleviez, nous devrons évidemment nous engager dans un système de licences stables et d'autorisations durables, pour la période qui court jusqu'à la fin du

Mme Colette Mélot. Monsieur le secrétaire d'État, le programme Erasmus+ ne fait pas partie de l'accord de commerce et de coopération négocié avec le Royaume-Uni. Cette volonté de dernière minute des Britanniques, nous ne pouvons que la regretter. Erasmus est l'un des symboles de la réussite européenne, c'est l'esprit de notre volonté de vivre ensemble. Depuis toujours, pour le Royaume-Uni, l'adhésion et la participation à l'Union européenne coûtent trop cher. Selon les Britanniques, Erasmus ne fait pas exception, particulièrement parce qu'ils accueillaient deux fois plus d'étudiants qu'ils n'en envoyaient dans le reste de l'Union européenne. On peut s'interroger légitimement

en juin 2018. Le résultat est sans appel : Erasmus est bénéfique pour les pays d'accueil. Plus intéressant encore, l'analyse conclut même que la balance économique est positive quand il y a plus de participants entrants que de participants sortants. Nous devrions encore voir des participants britanniques et européens bénéficier d'Erasmus+ jusqu'en 2023, le temps que la programmation 2014-2020 soit achevée. Mais la suite est incertaine, ce qui n'est pas sans morceler le Royaume-Uni lui-même. Le pays a décidé de développer son propre programme, le qui se veut concurrent, mais ne prévoirait pas l'accueil d'étudiants étrangers. Il concernerait 35 000 étudiants dès septembre 2021, pour un montant de 100 millions de livres. Les moyens alloués paraissent insuffisants en comparaison d'Erasmus+. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer sur les cas de l'Écosse et du Pays de Galles, qui ont manifesté leur intérêt pour continuer à participer au programme Erasmus+ ?

Nous pourrons avoir cette discussion bilatérale, mais je crois que c'est aujourd'hui aux Britanniques de préciser leurs intentions sur leur volonté ou non d'avoir une coopération universitaire avec nous. Dans le cadre de nos échanges bilatéraux, nous pourrons renforcer d'autres dispositifs spécifiques, comme celui des ou des

M. Guillaume Gontard. Monsieur le secrétaire d'État, quelques semaines après l'entrée en vigueur du Brexit, les inconnues et les questionnements sont encore légion. Parmi les causes de ce choix du peuple britannique, la question migratoire a joué un rôle important. Or, malgré les promesses des tenants de la sortie de l'Union européenne, le départ du Royaume-Uni ne signifie pas la fin de l'immigration sur son sol, car nous savons que les considérations légales pèsent peu face à la détermination des personnes migrantes. Les chiffres le prouvent : en 2020, plus de 9 500 passages ou tentatives de passage de la Manche ont été recensés, soit quatre fois plus qu'en 2019. Dans ce cadre, on déplore au moins six morts et trois disparus. La mise en oeuvre d'une politique migratoire orientée avant tout vers la sécurité humaine est donc absolument nécessaire, ma collègue Gisèle Jourda l'a parfaitement rappelé. L'accord dont nous discutons aujourd'hui passe pourtant sous silence l'ensemble de ces questions. Le règlement de Dublin ne s'appliquant plus au Royaume-Uni, l'incertitude prévaut quant à la gestion du renvoi de migrants illégaux vers l'Union européenne. Les conditions de regroupement familial pour les mineurs non accompagnés restent aussi en suspens. Quel est l'avenir des accords de Sandhurst de 2018 ? Faute d'un cadre de regroupement clair, ces mineurs prennent aujourd'hui de gros risques pour traverser la Manche. Cette nouvelle situation illustre davantage encore l'ineptie de la politique migratoire communautaire et ravive nos inquiétudes.

illégaux ? Entre le Royaume-Uni et la France, dans la mesure où la sécurisation massive des frontières ne dissuade personne de faire la traversée et ne fait que menacer des vies humaines, comment envisager une coopération future dans le respect des droits humains fondamentaux, notamment dans le cas de renvois systématiques vers la France ?

Dans les mois qui viennent, nous devrions, en lien avec nos partenaires européens, proposer au Royaume-Uni un accord dupliquant ou adaptant les règles de Dublin en matière de reconduite. Surtout, il conviendra de renforcer, au-delà de l'application de ces règles de reconduite, la coopération bilatérale qui nous unit au Royaume-Uni, pas seulement par les accords et protocoles que j'ai signalés, mais par des coopérations très opérationnelles. Je pense à celles que Priti Patel et Gérald Darmanin, les deux ministres de l'intérieur, ont conclues à la fin du mois de décembre, afin d'éviter les traversées de la Manche en renforçant nos moyens communs. Ces traversées ont quadruplé entre 2019 et 2020. En les empêchant, nous sommes à la fois plus efficaces dans la lutte contre l'immigration illégale et plus humains, parce que nous empêchons des drames. Nous avons refusé, comme le Royaume-Uni l'avait proposé, des interceptions en mer

M. Ludovic Haye. Monsieur le secrétaire d'État, nous avons pu observer ces dernières années un soutien actif et une contribution substantielle du Royaume-Uni à la mise en place d'une stratégie européenne de cybersécurité. L'expérience et l'expertise de ce pays dans le domaine de la cybersécurité sont largement respectées en Europe, le Royaume-Uni allant jusqu'à se positionner parfois en chef de file sur certains projets majeurs. Le Royaume-Uni a également permis une belle avancée en Europe dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, en fournissant du personnel et de l'expertise à Europol et à l'Agence européenne chargée de la Enfin, il a également efficacement travaillé avec les pays européens partageant sa vision, celle qui consiste à rechercher clairement la responsabilité de certaines grandes cyberattaques récentes, en encourageant d'autres pays à nommer les groupes responsables, parfois même les États commanditaires, mais aussi celle qui recherche une sanction

Monsieur le secrétaire d'État, bien que nous ayant déjà rassurés sur de nombreux points en commission, pourriez-vous nous dire si le Royaume-Uni a sollicité une invitation à participer à certaines activités de l'Enisa, notamment en matière de renforcement des capacités, connaissances et informations, ainsi que de sensibilisation et d'éducation, comme le prévoit l'accord ? échéant, des contacts ont-ils déjà pu être mis en place entre Londres et l'Enisa, afin d'évoquer les contours de cette future participation ? Qu'en sera-t-il de la participation britannique aux exercices de cybersécurité menés en Europe,

le Royaume-Uni au détriment de l'Union européenne, l'accord du 24 décembre comporte des garanties sur la concurrence loyale en matière de commerce et d'investissement. Je rappelle les deux principales, celle de non-régression en matière sociale, qui pourrait viser notamment le projet britannique de réforme du temps de travail, et celle concernant les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal. On ne peut que souscrire à ces

Le salaire mensuel minimum, par exemple, est de 312 euros seulement en Bulgarie. Le Parlement européen s'est d'ailleurs prononcé, le mois dernier, pour un salaire minimum européen. Ma question est simple, monsieur le secrétaire d'État : l'Union européenne est-elle prête à s'attaquer plus frontalement aux logiques fiscales

le risque de compétition existe. Déjà présent avant le Brexit, il demeure, et nous devons renforcer nos propres standards sociaux et fiscaux. C'est la bataille que nous avons engagée sur le travail détaché depuis 2017, avec une directive qui

à l'Union européenne, nous serons capables de les faire respecter dans le cadre de notre relation économique avec le Royaume-Uni. En matière fiscale, c'est sans doute plus difficile encore, car la règle de l'unanimité

Dans ce cadre, j'appelle tout particulièrement votre attention sur une thématique bien spécifique, celle des chambres de compensation. Créées après la crise des en 2008, ces institutions servent d'intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs de titres financiers. Sur un marché financier, toutes les opérations transitent par ces dernières, dont le rôle est de garantir la bonne tenue des transactions en assurant le règlement et la livraison des titres. Or la plupart de ces chambres, ou du moins les plus influentes, se trouvent au Royaume-Uni, désormais considéré comme un pays tiers.

Une éventuelle faillite d'une chambre de compensation londonienne aurait de lourdes conséquences financières et économiques pour l'Union européenne. Cette situation m'appelle à vous poser deux questions, monsieur

cet outil appelé « décision d'équivalence », qui reste toujours entre nos mains, de caractère provisoire et révocable. Pour les chambres de compensation en particulier, au regard de leur concentration au Royaume-Uni et de leur importance pour la continuité des services financiers, à la fin de l'année 2020, la Commission européenne avait donné une équivalence courant jusqu'à la mi-2022, permettant l'accès de nos opérateurs aux chambres de compensation britanniques. D'ici là, nous devons faire deux choses que vous évoquiez dans votre référence au règlement EMIR, monsieur

de l'Union européenne dans le domaine de la pêche s'était initialement développée avec l'ambition commune d'une pêche durable, innovante et compétitive. Elle était née de la volonté d'assurer la pérennité des pêcheries et de garantir des revenus et des emplois stables aux pêcheurs. Je souhaite à mon tour vous faire part de mes inquiétudes sur les négociations inachevées du volet pêche dans les accords du Brexit. Ce dernier affecte en effet plus de 600 navires français, dont les prises en eaux britanniques représentent 30 % du chiffre d'affaires. 92 % des pêcheurs britanniques auraient voté pour le Brexit. Compte tenu de leur insatisfaction et de leur volonté de retrouver une totale souveraineté sur leurs eaux, je crains que le secteur de la pêche ne soit sacrifié au profit d'autres domaines. Le saut dans l'inconnu que représente l'après-30 juin 2026 est préoccupant. Quelques semaines après l'entrée en vigueur de l'accord, nous percevons déjà une oscillation dans son application. Je pense ici au cas des îles anglo-normandes et à la perte de droits historiques séculaires applicables entre nos deux pays, qui nous donne un avant-goût de ce que pourraient devenir nos relations en termes de pêche à partir du 1 juillet 2026. Monsieur le secrétaire d'État, indépendamment de votre plan d'engagements à court terme, ma question est double. Après cette période de transition, ne doit-on pas redouter une diminution significative de l'accès de nos pêcheurs aux eaux britanniques ? À ce jour, quelle est l'avancée des négociations entre nos pays pour l'accès

le secrétaire d'État. Simplement, si j'ose dire, ce qui pèche pour ce secteur et son développement, c'est quand même l'incertitude de son devenir dans moins de six ans

ma question est relative aux droits des citoyens figurant dans l'accord de retrait, qu'il s'agisse des citoyens de l'Union européenne établis au Royaume-Uni ou des Britanniques établis dans l'Union européenne. Je pense en particulier aux Français qui vivent au Royaume-Uni. Selon le registre des Français établis hors de France, ils sont plus de 144 000. Toutefois, l'inscription au registre n'étant pas obligatoire, l'estimation réelle de la présence française au Royaume-Uni se situe plutôt entre 200 000 et 250 000 Français.

n'ont pas forcément accès à internet. Nous avons aussi au Royaume-Uni des compatriotes en situation fragile, qui n'ont pas accès à toutes les informations. Nous menons toutes les actions possibles pour les trouver et leur signaler cette date limite. Faut-il la repousser ? Honnêtement, je ne crois pas à ce stade, car ce serait prolonger l'incertitude.

La stupeur des premiers mois a été suivie par d'interminables négociations. Elles ont abouti, fort heureusement, à un accord de commerce et de coopération qui nous réunit aujourd'hui. Désormais, les ressortissants européens doivent faire face à cette nouvelle réalité et à ses nombreuses conséquences pour leur vie quotidienne. Si un grand nombre de difficultés persistent, l'un des sujets majeurs, qui cristallise les tensions, a trait au nouveau statut d'immigration, dont la demande doit impérativement être formulée avant le 30 juin 2021,

Une inquiétude persiste toutefois pour les personnes vulnérables, âgées ou isolées, qui ne maîtrisent pas forcément l'outil informatique.

Cette liberté des échanges, conjuguée à la proximité géographique du Royaume-Uni, à la taille de son économie et à son imbrication dans les chaînes de valeur du marché unique, rend l'exigence d'une concurrence équitable plus fondamentale que jamais pour ne pas saper la compétitivité de nos entreprises. Or la fiscalité, qui en est un levier fondamental, est largement absente des dispositions de l'accord, alors même que les autorités britanniques ont régulièrement affiché leur volonté de mener une stratégie fiscale agressive. Certes, un chapitre vient encadrer l'octroi des aides d'État, mais les autres pans de la fiscalité, notamment l'imposition sur les sociétés, n'entrent pas dans le champ d'application des mécanismes de résolution des différends et des mesures de rééquilibrage. Ils ne sont pas non plus concernés par le principe de non-régression convenu pour certaines normes sociales ou environnementales. Dans ces conditions, le spectre d'un dumping fiscal britannique semble désormais un danger bien réel. Monsieur le secrétaire

? La situation fiscale au Royaume-Uni sera-t-elle examinée au titre de la « liste noire des paradis fiscaux » de l'Union européenne ? Les dépendances de la Couronne- Jersey, Guernesey, île de Man -feront-elles l'objet d'une attention particulière ? Surtout, l'Europe et ses États membres vous paraissent-ils suffisamment armés, dans le cadre de cet accord, pour protéger leurs entreprises et répondre efficacement à un éventuel dumping fiscal britannique, qui viendrait s'ajouter aux difficultés déjà rencontrées à l'intérieur même du marché unique dans ce domaine ? La parole est à M. le secrétaire d'État. Monsieur le sénateur,

Nous n'avions jamais été confrontés à ce cas de figure depuis la création des communautés européennes, il y a près de soixante-dix ans. Nous étions probablement nombreux à penser que jamais un État ne quitterait l'Union. Le Royaume-Uni nous a pourtant donné tort, et l'Union européenne a su s'adapter en conséquence. Si nous devons nous réjouir d'être parvenus à trouver un terrain d'entente plutôt que d'avoir pris la voie d'un et des conséquences catastrophiques qui en auraient découlé, rappelons-nous toutefois que personne n'est gagnant avec cet accord. Il s'agissait simplement de recoller les pots cassés provoqués par la décision du Royaume-Uni. L'Union européenne a réussi à négocier un accord avec le moins possible de conséquences fâcheuses, mais il n'en reste pas moins que le départ du Royaume-Uni n'a que de mauvaises conséquences. Aucun bénéfice ne peut en être tiré par l'Union européenne comme par la France. Je ne citerai pas un à un les impacts du Brexit sur notre pays ; ils l'ont déjà été à maintes reprises. Mais je souhaite insister sur la nécessité et l'obligation qu'a le Gouvernement d'en réduire au maximum les effets. Maintenant qu'un accord a été conclu, il convient d'accompagner les acteurs économiques français face aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni du marché unique. Les entreprises françaises ont déjà été largement frappées par la crise sanitaire, nous ne pouvons pas les laisser subir également les effets du Brexit. Ma question, monsieur le secrétaire d'État, porte donc sur la façon dont le Gouvernement entend accompagner les entreprises françaises pour qu'elles s'adaptent aux nouvelles implications de cet accord et qu'elles en souffrent le moins possible. Le Gouvernement compte-t-il aider les entreprises qui perdront des parts de marché au Royaume-Uni face aux pays tiers ? Soutiendra-t-il les pêcheurs qui devront reverser une part de leurs prises et qui subiront en conséquence une perte de chiffre d'affaires ? Facilitera-t-il la délivrance de titres de séjour pour les saisonniers britanniques qui viennent travailler dans nos stations de ski ?

en prévoyant une absence de droits de douane et de contingents tarifaires sur les marchandises, l'accord conclu avec Londres a permis d'éviter la perturbation massive et immédiate des flux commerciaux qu'aurait inévitablement engendrée un. Le Le soulagement d'avoir évité le scénario du pire ne doit pas nous faire perdre de vue que le Brexit est avant tout, pour les autorités britanniques, le moyen de mettre en oeuvre leur projet de et de tourner leur regard vers d'autres régions du monde. Cette évolution aura des conséquences pour les producteurs du continent exportant outre-Manche. Le secteur du sucre, qui vient de connaître une année 2020 catastrophique, est à ce titre particulièrement concerné, car les producteurs français de betterave exportent 10 % de leur sucre et 15 % de leur éthanol au Royaume-Uni. Or celui-ci a décidé d'augmenter considérablement ses importations de sucre brut depuis les zones de production les plus compétitives au monde afin de les raffiner sur le territoire britannique. Le risque est donc grand de voir les parts de marché françaises s'y éroder avec le temps, mais aussi le sucre de betterave britannique, devenu excédentaire, se diriger à terme vers le marché européen. Monsieur le secrétaire d'État, avez-vous anticipé cette recomposition du commerce du sucre et prévu d'éventuelles mesures d'accompagnement ? L'accord de commerce et de coopération contient-il des clauses de sauvegarde, nous permettant de limiter les importations en cas de perturbation du marché intérieur ? La parole

de manière intelligente, un droit à la mobilité pour tous et, conséquemment, que tous les territoires devaient être couverts par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Néanmoins, certains territoires sont sans ressources ni modèle économique : l'égalité des territoires n'est pas assurée. Refusons des mobilités à deux vitesses et les fractures territoriales et sociales ainsi provoquées.

Les mobilités s'organisent d'une manière très différente entre les espaces denses et peu denses. Dans un cas, la massification est possible- tramways, métros, TGV, transports en commun en site propre, etc. -, les

D'ailleurs, certains des intervenants et experts que nous avons auditionnés définissent ces territoires peu denses comme étant ceux où il n'y a que la voiture pour se déplacer ou encore ceux dans lesquels le transport coûte cher dans le budget des ménages. La situation est radicalement différente en fonction de la situation dans laquelle on se trouve : dans le rural polarisé autour d'un centre, l'organisation sera différente

effectuer moins de déplacements subis grâce à un bon positionnement des services par rapport à l'habitat ? Cela nécessite des politiques audacieuses d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la prise en compte de la gestion des temps, et donc une bonne échelle de gouvernance, proche des bassins de mobilité

La première : utiliser l'existant et le renforcer, qu'il s'agisse des petites lignes ferroviaires ou des services réguliers de cars interurbains, le cas échéant en organisant des rabattements, en les modernisant,

où la puissance politique n'interviendrait qu' ; par conséquent, les évolutions proviendraient des ruptures technologiques et de la logique de marché. La décarbonation serait le fait des véhicules électriques.

Monsieur le secrétaire d'État, nous avons besoin d'un modèle économique pour financer cette politique publique maintenant imposée. C'est une question d'égalité intervention en citant l'un des meilleurs spécialistes des mobilités, Gilles Dansart : « Il ne s'agit pas non plus d'opposer la mobilité individuelle aux transports collectifs, ce qui empoisonne le débat et ralentit les mutations. En effet, une mobilité moderne et décarbonée est possible, y compris pour les espaces peu denses, en s'appuyant sur le triptyque proximité-intermodalité-accessibilité pour lutter contre les mobilités à deux vitesses entre territoires urbains bien pourvus et espaces peu denses déséquipés et sans autre solution que le recours à la voiture. Il s'agit donc bien de lutter contre les fractures territoriales et sociales actuelles.

présidente, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, permettez-moi d'emblée de remercier la délégation sénatoriale à la prospective, en particulier son rapporteur, Olivier Jacquin, d'avoir demandé l'organisation de ce débat.

la ruralité. La mobilité est l'un des grands enjeux de l'attractivité des territoires ruraux ; elle constitue à ce titre un volet important de l'agenda rural que je suis chargé de mettre en oeuvre

Les espaces peu denses, dans lesquels vivent un tiers des habitants du pays, nécessitent une politique de transport adaptée à cette réalité qui est bien différente de celle que connaissent les citadins. Il serait vain et contreproductif de désigner la voiture individuelle comme une ennemie à éradiquer. Pour autant, tout l'enjeu de nos politiques, c'est de ne pas se résigner à ce que certains ont nommé « l'autosolisme », un néologisme pas très élégant. Il s'agit non pas d'éliminer la voiture, mais d'en favoriser un usage plus collectif, ainsi que les alternatives. L'enjeu est de réduire L'enjeu est de réduire la dépendance à la voiture, car elle est source de fragilités et d'inégalités. Elle est d'abord source de fragilités pour les territoires qui perdent en attractivité faute d'une offre de mobilité suffisante et adaptée.

C'est d'ailleurs tout l'objet de la loi d'orientation des mobilités (LOM) qui prévoit des investissements sans précédent et fixe comme priorité les transports du quotidien. Il s'agit de la loi la plus importante sur ce sujet depuis la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI), adoptée en 1982, et la loi relative La LOM prévoit de couvrir l'ensemble du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité, une AOM. Désormais, et c'est un acquis important de ce quinquennat, il n'y aura plus de zone blanche en ce qui concerne la mobilité. Les communautés de communes sont ainsi encouragées à délibérer pour se saisir de cette compétence avant le 31 de ce mois ; à défaut, la région assurera ce rôle d'AOM locale pour déployer une offre de proximité au niveau des bassins de mobilité. Sur ce sujet, je veux rappeler la responsabilité des collectivités locales dans l'exercice de cette compétence. En voyage officiel la semaine dernière, j'ai pu constater les tensions entre EPCI et régions sur la définition et le financement des transports de proximité. L'esprit de la LOM est bien de construire un maillage territorial et une complémentarité entre les services de mobilité offerts à tous les échelons- local, régional et national. Il ne s'agit pas, par exemple, comme il nous a été rapporté à l'occasion de ce déplacement, d'appeler les intercommunalités rurales à cofinancer les services ferroviaires régionaux au motif qu'elles en bénéficient. Le législateur a voulu que les territoires soient en première ligne pour définir leurs offres de mobilité au plus près des besoins. Pour autant, l'État ne livre pas les territoires à eux-mêmes. Ainsi, le Gouvernement a développé la démarche France Mobilités, bras opérationnel de la LOM elle a pour mission d'identifier les solutions de mobilité, d'en faciliter l'expérimentation, de contribuer à leur montée en puissance et de les déployer largement, lorsque c'est possible. Je me réjouis d'ailleurs de l'engouement que j'observe sur les appels à manifestation d'intérêt de France Mobilités mobilités durables (Tenmod), nous avons déjà financé 92 projets pour un total de 6,7 millions d'euros, tous en zone peu dense. Nous croyons aussi à toutes les formes de socialisation de la voiture, comme le covoiturage ou l'autopartage. Les différents appels à projets permettent de soutenir, en lien avec les collectivités, l'expérimentation de nouvelles solutions de plateforme de mobilité permettant, grâce à l'intelligence artificielle, de renouveler les offres de covoiturage ou de transport à la demande développées par un tissu de start-up innovantes.

Au-delà de cette incitation financière bienvenue, le Gouvernement a mis en oeuvre plusieurs outils budgétaires pour redynamiser le vélo, un mode de transport pratique, écologique, économique et, accessoirement, bon pour la santé ... Le vélo a aussi sa place en zone peu dense, dès lors bien évidemment que la géomorphologie le permet. Nous avons par exemple doté de 215 millions d'euros le fonds national Mobilités actives pour soutenir les projets structurants des collectivités qui prévoient de créer des axes cyclables sécurisés. Ce sont ainsi 119 millions qui ont été alloués à 259 projets en milieu rural. De plus, le coup de pouce « vélo », doté de 200 millions d'euros, a permis d'aider tous ceux qui ont souhaité réparer leur vélo pour en faire leur moyen de déplacement quotidien. Parallèlement, nous investissons sur le ferroviaire. Conformément à la priorité affichée dès le début du quinquennat en faveur des transports du quotidien et du réseau existant, le Gouvernement a décidé d'investir massivement dans le réseau ferroviaire. Les besoins d'investissements pour la régénération de ces lignes se chiffrent à 7,5 milliards d'euros pour la décennie qui s'ouvre. Près de 1,5 milliard d'euros sont financés dès la période 2020-2022, 2020-2022, l'État apportant plus de 500 millions, dont 300 millions dans le cadre du plan de relance. Cet investissement conjoint avec les régions devra se poursuivre tout au long de la décennie pour atteindre nos objectifs. La remise à niveau de nos infrastructures ferroviaires est une politique de long terme. Je soutiens par ailleurs le redéploiement d'une offre attractive de trains Intercités de jour et de nuit qui permettra des relations entre territoires en dehors du réseau à grande vitesse. Il nous faut aussi proposer une offre de transport attractive alternative à la voiture pour ceux qui, à la suite du confinement, ont choisi de s'éloigner des grandes villes pour s'installer dans la ruralité et y télétravailler. Il nous faudra également faire en sorte d'améliorer l'information des voyageurs au niveau national pour garantir à tous l'accès à l'information sur l'ensemble des offres disponibles, et ce jusqu'au dernier kilomètre. Cette information est trop morcelée entre différents sites. Ces politiques, si elles ne montrent pas encore tous leurs effets,

de garantir l'équité et la cohésion des territoires. Voilà ce que je tenais à vous dire en prélude à ce débat. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous allons maintenant Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.

contre seulement 1,3 personne par véhicule individuel, permet de multiplier les offres de mobilité grâce à une certaine flexibilité et à une convivialité reconnue. Dans les zones moins denses, où les solutions de mobilité sont réduites, le partage du quotidien nécessite de la réactivité et une technologie développée pour effectuer une réservation et une mise en relation des populations intéressées. Ces initiatives s'articulent autour de deux principes : le covoiturage et le copartage. mode de transport, il s'agit de mettre en relation des citoyens effectuant des trajets courts. Le second se caractérise par le partage d'un véhicule entre plusieurs personnes. Une solution innovante de copartage a d'ailleurs vu le jour dans une communauté de communes de mon département, plus précisément Une expérimentation a été mise en place pour accompagner le prêt de véhicules de personnes qui ne les utilisent plus, souvent du fait de leur âge, au profit de personnes qui n'en ont pas. Cette coordination solidaire permet à chacun de se rendre chez le médecin, dans un service public ou, encore, dans les commerces de proximité. Ces services doivent être qualifiés de services publics. Aussi, il convient d'engager l'État dans une réflexion afin de proposer une coordination de différents services de transport. Cette application pourrait être accessible à tous, y compris au sein des maisons France Services. d'État, le Gouvernement envisage-t-il d'harmoniser l'ensemble de ces initiatives ? Comptez-vous mettre en place rapidement un budget pour travailler sur ces moyens d'avenir ? Accompagnerez-vous les zones rurales dans leur transition pour laquelle les particuliers sont l'indispensable maillon ?

comme vous le soulignez, ou sur la mise à disposition de véhicules. De nombreux montages peuvent exister sur les territoires. Aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui le permet et l'encourage. La loi d'orientation des mobilités a créé très clairement une compétence mobilités solidaires, qui impose la mise en place systématique, à l'échelle de chaque bassin de mobilité, d'un plan d'action commun en faveur des mobilités solidaires pour rendre nos services plus inclusifs par la tarification, l'information et l'accompagnement des personnes qui en ont besoin. Il s'agit de mettre en place de nouvelles solutions de transport d'utilité sociale, des garages solidaires, du covoiturage solidaire ou encore le prêt de véhicule.

imposé nationalement, mais de favoriser l'émergence de services qui sont adaptés aux réalités de chaque territoire. Dans cette mise en oeuvre d'une politique décentralisée, l'État entend être un facilitateur. C'est le sens, d'ailleurs, de la création de France Mobilités,

et le secteur des transports en produit une part importante. La stratégie nationale bas-carbone vise une réduction de 28 % des émissions de ce secteur d'ici à 2030, c'est-à-dire dans seulement neuf ans. Les zones peu denses sont révélatrices non seulement de notre retard en la matière, mais également, et je le regrette, du désintérêt porté à nos territoires ruraux : abandon des petites lignes, faiblesse des investissements, report multimodal en berne. Ce manque d'action se fait non seulement au détriment de notre avenir climatique, mais aussi au mépris de la moitié de la population française, qui vit et habite dans des territoires à faible densité et n'a souvent pas d'autre solution que la voiture. Ce rapport le montre, nous sommes face à un véritable défi de diversification des mobilités. Il pointe aussi les dérives qui s'installent : ainsi, pendant les trente dernières années, la proportion des déplacements effectués à pied pour se rendre à l'école ou au collège est passée de 52 % à 32 % ; dans le même temps, la proportion des déplacements à vélo a diminué de plus de moitié, passant de 7,5 % à 3,3 %. Il y a là un vrai sujet Le plan Vélo, lancé en 2020, n'est malheureusement pas à la hauteur des enjeux. L'aménagement des infrastructures doit être un levier de cette politique, car un des freins est bien lié à la sécurité, notamment pour les parents. pour les parents. Or les aménagements de voirie restent coûteux et les départements, les communes n'ont souvent pas les finances nécessaires pour envisager un plan ambitieux de construction de cheminements doux, en particulier des pistes cyclables. Cette question du financement est cruciale et déterminera l'atteinte ou non de nos objectifs environnementaux. quand et comment allez-vous réellement permettre l'essor d'une solution alternative au « tout-voiture » dans nos territoires peu denses ? Quelles solutions envisagez-vous pour sécuriser, notamment, les trajets pour se rendre à l'école et généraliser la marche à pied ou la circulation à vélo, ce qui est excellent pour la santé, vertueux pour l'environnement et bon pour le porte-monnaie des parents

qui a un fort potentiel, dans les zones peu denses comme dans les zones urbaines. Quel que soit le type de territoire, entre 30 % et 50 % des déplacements font entre 1 kilomètre et 5 kilomètres. Les collectivités locales se sont vraiment emparées de ce mode de transport pour déployer des politiques publiques de soutien local. Je tiens à saluer cet engagement, qui est nécessaire. un premier enjeu consiste à multiplier les itinéraires cyclables sécurisés. C'est ce que finance précisément le Fonds mobilités actives, qui a été mis en place dès 2019. Nous venons d'annoncer la liste des lauréats de la troisième édition. Au total, ce sont 533 projets qui ont été soutenus, pour 215 millions d'euros de subventions. de subventions. La moitié est en zone peu dense et en outre-mer, avec des taux de subvention bonifiés qui vont de 40 % à 70 %. D'autres financements sont accessibles aux collectivités, avec la la dotation régionale d'investissement, qui est déployée à l'occasion du plan de relance, et des aides qui sont recensées sur la plateforme aides.francemobilités.fr. Il y a également

D'autres outils doivent être développés par les territoires : le stationnement, l'aide à l'achat, la location. Là encore, l'État prévoit des mesures d'accompagnement. Enfin, chaque territoire est invité à faire la promotion du vélo auprès des habitants et des employeurs. Je les invite tous à se joindre à l'opération « Mai à vélo » pour donner envie de vélo. Il s'agit

particulièrement à ce que les financements qui vous ont été promis soient bien évidemment inscrits. Je ne vais pas vous faire une longue litanie des financements qui ont été prévus dans le Grand Est, notamment sur l'année 2020. Cet effort va se poursuivre en 2021, avec encore de de nouveaux financements, pour près de 15 millions d'euros, sur les petites lignes du Grand Est. Nous n'abandonnerons pas ces lignes et nous surveillerons attentivement les problématiques de la desserte fine des territoires que la SNCF doit mettre en place., nous exigerons que l'on revienne à la situation, qui était plus favorable que celles que vous connaissez

le changement climatique. Je suis persuadée que cela passe par la décarbonation de nos déplacements, le transport collectif et la multimodalité. Le biogaz, l'électricité, l'hydrogène et toutes sortes de mobilités douces sont primordiaux, tout comme l'innovation industrielle française dans ces secteurs. La clé de réussite se trouve dans le développement des infrastructures et dans un maillage territorial répondant aux nécessités de l'aménagement et de la transition écologique. Dans notre région Grand Est, nous expérimentons la multimodalité. Si j'appelle de mes voeux la décarbonation du secteur routier, je crois aussi que le transport des marchandises doit s'appréhender différemment. C'est pourquoi je soutiens l'expérimentation du train à hydrogène et la mise à grand gabarit du canal de la Seine jusqu'à Nogent-sur-Seine. Ce projet prouve que le report modal est très pertinent. Il relève d'une modernisation plus large des infrastructures, où les échanges entre territoires le fluvial deviennent une réalité. C'est le genre de cercle vertueux dont la France a besoin. Les idées et les innovations dans le domaine de la mobilité sont nombreuses et émanent souvent des acteurs locaux. La solution viendra des territoires et sera déterminante pour notre souveraineté industrielle. Monsieur le secrétaire d'État, tout ce que je viens d'évoquer requiert des efforts financiers financiers et des capitaux énormes. Les secteurs public et privé, les échelons national et locaux doivent s'associer pour réussir cette relance. Quelles sont vos solutions, hors plan de relance, pour mobiliser ces moyens à court et moyen termes, pour le bénéfice de nos territoires, surtout les moins denses ? La parole

Ensemble, ils financent toutes les actions qui sont engagées par l'État pour les modes routier, ferroviaire, fluvial et portuaire. Dans le cadre de la loi

Ce montant comprend la trajectoire financière inscrite dans la loi d'orientation des mobilités, que nous respectons donc, à laquelle s'ajoute l'engagement financier de l'État sur le canal Seine-Nord Europe. Conformément aux principes définis dans la LOM, la priorité est donnée à la maintenance des réseaux et au report modal. S'agissant spécifiquement de la poursuite de la mise à grand gabarit de la Seine, à travers le projet de canal entre Bray et Nogent-sur-Seine, je me réjouis de votre soutien. Ce projet de développement du réseau fluvial, dont le financement est projeté à partir de 2028

Comme vous le soulignez, c'est un investissement qui doit vraiment stimuler le développement économique local en bénéficiant aux chargeurs, aux industriels, dans un contexte de croissance continue

et 1,5 million de tonnes aujourd'hui. Ce trafic additionnel correspond pour l'essentiel à un report modal, que vous appelez de vos voeux, par rapport à la route. Il a été estimé que 27 000 trajets de camions seront ainsi évités chaque année. Madame

de nouvelles mobilités, telles que la mobilité hydrogène. C'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi en vue de créer des fonds souverains régionaux, qui seraient abondés partiellement par la sur-épargne des Français pendant la crise sanitaire. Je souhaite que nous puissions débattre prochainement de cet instrument

met en valeur, parmi la palette d'alternatives à la voiture, le potentiel du vélo, qu'il s'agisse du vélo classique, du vélo électrique, mais aussi des innovations de type tricycle caréné, en devenir. Ces dernières années, et encore plus ces tout derniers mois, nous avons assisté à un développement du vélo et à une avancée nette dans l'opinion. Même si cette progression récente a été plus marquée en ville, elle a aussi concerné la campagne. Le rapport de notre collègue autres mérites, celui de démonter cette idée reçue de l'inaptitude supposée du vélo à se faire sa place à la campagne pour les mobilités du quotidien. Le rapport pointe cependant les difficultés spécifiques au développement du vélo en zone peu dense : la nécessité d'un véritable « système vélo », intégrant des aménagements de voiries, d'autant plus indispensables que le différentiel de vitesse avec les autres usagers est bien plus marqué qu'en zone urbaine, des possibilités sécurisées de stationnement et de bonnes conditions de rabattement et d'embarquement vers

ce que l'Eurométropole de Strasbourg à elle seule compte investir lors de cette mandature en infrastructures cyclables. Monsieur le secrétaire d'État, au-delà des appels à projets, le Gouvernement envisage-t-il une réelle montée en puissance pour généraliser les aménagements cyclables de voiries, et, plus globalement, pour massifier de nouvelles dynamiques de report sur les mobilités actives ? Si oui, quelles solutions avancez-vous ?

et nous mettons en oeuvre des moyens considérables pour y arriver. Il s'agit de moyens d'ingénierie, d'une part, parce que le premier levier pour encourager la pratique du vélo, c'est quand même d'aménager des pistes cyclables sécurisées. Nous en parlions à l'instant. les collectivités auront besoin d'un appui technique important et fiable, dont elles ne disposent pas toujours. J'ai créé des réseaux de voies vertes et de véloroute sur un secteur, et je vous prie de croire que nous avons rencontré des difficultés pour bénéficier d'ingénierie en la matière.

et plus particulièrement sur un territoire bien plus connu aujourd'hui pour son apport à notre excellence agroalimentaire et brassicole que pour les questions de mobilité : je veux ici parler des Flandres, plus précisément de la communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI). Son tout jeune président, Valentin Belleval, s'est saisi, dès son élection, voilà quelques mois, de la problématique des mobilités sur son territoire, et il est en passe, avec ses collègues de la CCFI, de prendre la compétence mobilités au 31 mars. Voilà un territoire rural et périurbain, composé de 50 communes réparties sur un territoire de 630 kilomètres carrés, avec environ 105 000 habitants pour lesquels les déplacements quotidiens portent sur des distances importantes, souvent supérieures à 30 kilomètres. L'usage de la voiture personnelle y est prédominant, faute, à ce jour, de solutions alternatives efficaces. type de territoire, la faculté de se déplacer est un enjeu capital, car elle conditionne l'accès aux différents services, de santé, d'éducation, de consommation, et également à l'emploi. L'exigence de mobilité est devenue une norme et celles et ceux qui ne peuvent y répondre voient leurs capacités d'intégration sociale et professionnelle minorées. Pourtant, cette communauté de communes dispose d'atouts non négligeables, avec une collectivité déjà fortement impliquée dans les questions de mobilité, un réseau ferré très développé et un réseau interurbain complémentaire. Néanmoins, ce territoire a aussi ses faiblesses : six de ses communes sont des zones blanches de mobilité ; le réseau interurbain est à fort usage scolaire et les zones d'emploi sont difficiles à desservir.

possède une longue frontière avec la Belgique, où sont recensées de nombreuses petites communes, elle aussi en zone blanche, qui souhaitent bénéficier des atouts de la ville centre, Hazebrouck, notamment pour la desserte ferroviaire. La question des mobilités en espaces peu denses se joue non pas à l'horizon de 2040, mais dès aujourd'hui sur ce territoire, comme sur bien d'autres dans notre pays. Ma question sera donc simple : quelles sont les possibilités qui s'offrent à la CCFI, mais aussi, au-delà, à tous nos territoires transfrontaliers, pour favoriser le transport dans les zones peu denses de chaque côté de la frontière avec la prise de compétence mobilités ? La

vouloir prendre au travers de votre intercommunalité, est un choix fort. Il faut bien comprendre que les évolutions de gouvernance portées par la LOM sont fondamentales, au sens où elles ne réduisent pas les enjeux de mobilité aux seules zones urbaines. Elles concernent également des zones peu denses. En encourageant les territoires ruraux à se saisir de la compétence, en instaurant un dialogue systématique à l'échelle du bassin de vie entre acteurs de la mobilité, la LOM permet de mettre à l'agenda politique et technique des problématiques des territoires ruraux, mobilité (AOM) seront les porte-parole auprès des territoires limitrophes et des régions, et de faire en sorte que les politiques de mobilités soient décloisonnées pour assurer une meilleure intermodalité. Ces contrats de mobilité, qui pourront déboucher sur des structures de gouvernance, sont des outils fédérateurs pour construire un système de mobilité plus intégré et plus cohérent au regard des pratiques quotidiennes des habitants des territoires,

dont le Parlement devrait être saisi prochainement, va être un véhicule législatif pertinent pour renforcer les capacités des collectivités à s'entendre avec les autorités locales de nos voisins pour conforter cette coopération territoriale, qu'il s'agisse de mobilités, mais aussi d'autres sujets extrêmement importants. Je pense notamment au domaine de la santé.

ainsi les mobilités. Des siècles plus tard, il est nécessaire de continuer à nourrir la réflexion sur leur évolution, ce à quoi le rapporteur a entendu contribuer en se projetant dans l'avenir à l'aune des évolutions technologiques et sociétales. Le rapport dresse des constats indéniables, que je partage, pointe le risque d'un progrès à deux vitesses entre les territoires urbains et ruraux, et dessine divers scénarios susceptibles de se réaliser. La crise du covid-19 est passée par là, venant bousculer notre quotidien et nos certitudes dans nos relations avec les autres, nos loisirs, notre manière d'étudier, de travailler, de consommer, de consulter un professionnel de santé et, partant, de nous déplacer. Alors que certaines discussions se bornaient aux grands chantiers d'infrastructures routières, les data sont venues bousculer nos habitudes et pallier et pallier les contraintes des mesures sanitaires qui nous sont imposées. Le rapport souligne précisément ces transformations, avançant que nous pourrions entrer dans une nouvelle ère de la « démobilité », où nous verrions se réduire les mobilités subies au profit des mobilités choisies. À l'heure du digital et à l'expérience de la crise du covid-19, ne vaut-il pas mieux faire transiter les données les réseaux plutôt que les hommes sur les routes ? N'est-il pas préférable de traiter la cause des déplacements plutôt que leurs conséquences ? La « démobilité » n'est-elle pas à considérer comme un levier de développement pour les territoires ruraux et peu denses ? Pour permettre à ces territoires de se réinventer, le développement de la couverture numérique en très haut débit, à l'instar du déploiement de la fibre optique en région Grand Est, est un préalable, tout comme l'accompagnement des populations vers l'accès aux services digitaux. J'ai bien conscience de prendre un peu le contre-pied du rapport, mais, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous assurer que mobilité et « démobilité » sont bien prises en compte par le Gouvernement dans une vision d'avenir de nos territoires ? Comment, et avec quels moyens, comptez-vous intégrer cette notion de « démobilité » dans la mobilité ? La parole est à M. le secrétaire

Aujourd'hui, près des trois quarts des télétravailleurs occasionnels souhaitent pouvoir télétravailler davantage ; ce phénomène est appelé à s'intensifier. On constate aussi que de nombreux Français quittent les grands centres urbains et donnent ainsi une aura de précurseur au président Pompidou, qui écrivait ceci dans une lettre à Jacques Chaban-Delmas, en 1970 La vie moderne, dans son cadre de béton, de bitume et de néon créera de plus en plus chez tous un besoin d'évasion, de nature et de beauté. » Ce phénomène est aussi rendu possible par l'investissement sans précédent réalisé par ce gouvernement, notamment dans le cadre du New Deal mobile, pour résorber les zones blanches téléphoniques. Par ailleurs, les Français qui pratiquent l'exode rurbain ne vont pas pour autant cesser totalement de se rendre sur un lieu de travail. Probablement, une ou deux fois par semaine, ils devront prendre des transports ; il est donc nécessaire de poursuivre le maillage territorial en matière d'offre de mobilité, de manière à répondre aux besoins des habitants ruraux et à leur offrir une alternative au tout-voiture.

par la fin des zones blanches de la mobilité, puisque chaque territoire sera désormais couvert par une autorité compétente pour organiser une offre locale. C'est vraiment en ce sens que le déploiement des technologies et du numérique contribue au développement de services de mobilité partout, pour tous et pour tout,

Très bien ! En même temps, la LOM pousse les intercommunalités à se saisir de la compétence mobilités et laisse le soin aux régions dites chef de file d'assumer la compétence là où les intercommunalités ne le feraient pas. Pardonnez-moi, mais ma grand-mère aurait appelé cela l'art de gérer les restes. Or il n'y a rien de plus compliqué à faire, du point de vue économique, que de gérer ce qui reste.

Il eût été bon qu'on en tirât quelques enseignements ! Or, aujourd'hui, quand je défends des petites lignes ferroviaires, des lignes dites d'aménagement, ou de desserte fine du territoire- je crois que c'est ainsi qu'on les -, on me rétorque que nous sommes en train de désendetter la SNCF. Certes, mais on le fait en lui interdisant d'investir, ce qui revient à lui faire payer le prix de son désendettement.

en matière de nouveaux modes de déplacement. S'il reste nécessaire d'étudier la question des mobilités dans les espaces peu denses, c'est bien parce qu'elle est fondamentalement préoccupante, tant les écarts entre villes et campagnes se creusent. Le rapport de notre délégation à la prospective saisit avec justesse les domaines pour lesquels le monde rural peut légitimement s'inquiéter concernant ses possibilités de développement d'ici à 2040. Cependant, j'ose imaginer que nous n'en serons pas réduits à explorer des modes de déplacement alternatifs à la voiture par défaut ou par obligation ; je ne saurais croire que ce serait la seule chose qu'il nous reste à espérer Monsieur le secrétaire d'État, vous savez mieux que quiconque qu'il reste des fractures territoriales à réduire ; il reste même des frontières à franchir ! Je copréside depuis cinq ans le comité de massif du Jura, qui s'étend sur quatre départements : l'Ain, le Jura, le Doubs et le Territoire de Belfort. Unanimement, les 57 membres du comité réclament une voie rapide reliant le Jura à Lausanne. En effet, chaque jour, plus de 40 000 frontaliers empruntent des routes de misère pour aller travailler. Le covoiturage ou le bus ne peuvent résoudre notre manque flagrant d'infrastructures. Depuis plus de trente ans, élus français et suisses de l'arc jurassien demandent une voie rapide, mais puisqu'ils ne sont pas nombreux- autrement dit, peu denses ! -, les gouvernements successifs les ont ignorés. Monsieur le secrétaire d'État, est-ce donc une fatalité ? Les territoires mal desservis sont-ils condamnés à l'immobilisme, ou bien pouvons-nous compter sur le montagnard que vous êtes pour soutenir notre projet et franchir le massif du Jura ?

Je tiens, madame la sénatrice, à réaffirmer l'engagement de l'État pour améliorer les conditions de sécurité et de circulation sur les routes nationales dans le Jura.

passe par Genève, en empruntant l'autoroute A40. Si le projet de liaison routière Poligny et Vallorbe n'a pas été retenu à ce jour parmi les priorités de l'État, son opportunité pourra être à nouveau discutée dans le cadre de l'élaboration de la prochaine contractualisation avec la région Bourgogne-Franche-Comté. L'État reste par ailleurs soucieux du niveau de service qui est offert aux usagers du réseau routier national ; il est donc naturellement prêt à poursuivre l'amélioration des itinéraires existants, notamment du point de vue de la sécurité routière. Nous nous montrerons ouverts aux sollicitations des collectivités territoriales dans la perspective des possibilités qu'offrira sans doute le

Reste à savoir si tous les outils offerts par cette loi pourront effectivement être utilisés par les acteurs locaux. En effet, leur mise en oeuvre dépend beaucoup de l'importance de l'importance des moyens financiers mis à disposition des collectivités et, notamment, de leur capacité à lever le versement mobilité auprès des entreprises. Certaines collectivités ne disposent pas de bases fiscales suffisantes sur leur territoire et risquent de se retrouver démunies, leurs ressources s'avérant trop faibles pour pouvoir mettre en place des solutions de mobilités. Par ailleurs, l'émergence de pratiques innovantes est parfois contrariée par le manque de compétences et d'expertises disponibles pour les collectivités. S'il existe en théorie une palette de solutions alternatives à la voiture individuelle dans les zones peu denses, les difficultés techniques et juridiques rencontrées dans leur mise en place et leur fonctionnement

un accompagnement sur mesure des projets qui n'entrent pas dans les deux précédentes catégories. L'intervention de cette agence repose un certain nombre de principes, mais surtout sur une méthode de déconcentration au niveau des préfets, qui en sont les délégués territoriaux,

Mme Else Joseph. Monsieur le secrétaire d'État, l'avenir des mobilités est un défi pour nos territoires. Les mobilités seront notamment la clé de la sortie de crise, que nous espérons proche. Sans une offre polyvalente en la matière, nous ne pourrons envisager de reprise économique et sociale. notre délégation à la prospective, que je salue, la combinaison des modes constitue la solution. Il ne faut pas opposer les mobilités classiques aux mobilités nouvelles, mais les développer et les améliorer ensemble, car tout frein apporté à une mobilité rejaillit inévitablement sur une autre.

Le vélotourisme peut être une solution pour l'attractivité de nos territoires : c'est le cas avec cette véloroute EuroVelo 19. L'automobile reste indispensable, car elle est souvent le seul moyen d'accéder à nos centres-bourgs et aux services. Je ne me résous pas au phénomène d'assignation territoriale dû au fait que 20 % des personnes adultes vivant en zone peu dense ne disposent pas de voiture ! Réfléchissons à ses usages collectifs, comme l'autopartage, que nous pratiquons depuis deux ans.

prend sa part tout en donnant cette responsabilité aux collectivités, qui sont les mieux à même d'adapter efficacement les politiques publiques à leur territoire, comme vous le faites d'ailleurs dans votre département. Toutes les bonnes volontés convergent pour développer de vraies offres de mobilité

Il est ainsi noté, à la page 54 de ce rapport : « Avec le développement des livraisons, la logistique du dernier kilomètre est plus compliquée et coûteuse à développer lorsque les distances entre plusieurs clients sont particulièrement longues à parcourir. Aucun marché de la livraison ne pourra se développer sans organisation, sans coordination entre acteurs. Des acteurs déjà présents sur le territoire, comme La Poste, pourraient être incités encore plus à se saisir de cette question pour développer un panel de services de livraison aux habitants. » Le rapport souligne également que l'absence de service de livraison dans les espaces peu denses pourrait pénaliser l'attractivité de ces territoires. Aussi, les plans de mobilité rurale, bien qu'orientés principalement aujourd'hui vers la mobilité des personnes, devraient s'intéresser aussi à la dimension logistique et aux flux qui en résultent, comme cela est proposé dans la LOM. Monsieur le secrétaire

avec la fermeture de ses bureaux, la réduction des amplitudes d'ouverture et le nouveau concept de facteur guichetier. Alors, sur quels leviers doit-on agir pour que La Poste, qui est déjà présente sur ce segment de service, en amont, avec « Ma ville mon shopping », comme en aval, avec GeoPost, avec GeoPost, puisse mieux se déployer dans le domaine de la logistique si vital pour nos territoires ruraux ? Il faudrait que cela se fasse, bien évidemment, en garantissant une égalité de traitement territorial dans le niveau de la qualité du service apporté.

nombreuses, compte tenu des délais de livraison promis par les sites de vente en ligne. Cette situation engendre une pollution atmosphérique accrue ; de surcroît, ce type de livraison n'est pas rentable pour La Poste, ce qui met d'ailleurs en péril son modèle économique de livraison de colis en zone peu dense. Il convient donc de mutualiser les livraisons afin de maximiser le taux de chargement des véhicules qui assurent ces rotations. Une première solution, que nous mettons déjà en oeuvre, consiste à inciter La Poste et les sites de vente en ligne à se coordonner pour regrouper les colis. Quitte à allonger les délais d'attente, cette solution permettrait d'assurer un meilleur remplissage et de rendre l'activité plus soutenable financièrement. Une solution complémentaire serait la mise en place de plateformes de mutualisation des livraisons qui rassembleraient des acteurs locaux qui réalisent des livraisons- La Poste, par exemple -et un certain nombre d'artisans qui les font également. la plateforme numérique pourrait être la collectivité territoriale, La Poste, ou un acteur privé. La logistique du dernier kilomètre, qui est aussi importante pour les personnes que pour les marchandises, fait d'ailleurs partie des thèmes qui sont mis en avant dans la démarche « Action coeur de ville » coeur de ville » que le ministère de la cohésion des territoires met en oeuvre pour soutenir l'attractivité des villes moyennes. Le Cerema a également lancé un programme d'études pour élaborer de nouvelles solutions permettant aux collectivités de mieux gérer ces nouveaux flux logistiques.

était l'ambition de la LOM : rayer de la carte de France les zones blanches. Dans ce cadre, les transports ferrés connectés aux services de rabattement font figure de solution idéale. Pourtant, la question des dessertes fines ferrées rurales reste toujours soumise à un paradoxe et à une équation difficile.

à l'échelle hexagonale, la question reste entière. En 2021, les crédits consacrés aux lignes de desserte fine du territoire s'élèvent à 620 millions d'euros. Si cet effort peut être salué, il reste bien inférieur aux besoins identifiés

Plus largement, cette question pose également la pérennité du dispositif de soutien à toutes les infrastructures de transport. Ce soutien n'est pas assuré au-delà du plan de relance. Du fait de l'absence des mandats transports

puisqu'il apporte plus de 500 millions d'euros sur ces trois années, dont 300 millions au titre du plan de relance. Ces financements se font dans le cadre d'investissements de régénération qui approchent 1,5 milliard d'euros, en incluant les financements des régions et de SNCF Réseau.

les protocoles d'accord avec les régions, qui sont dans leur majorité signés ou en passe de l'être, sont précisément le cadre de notre engagement commun à pérenniser ces lignes. La première garantie est le recensement exhaustif des besoins et des modalités de financement, ligne par ligne, financeur par financeur. Nul acteur ne pourra donc s'exonérer, qu'il s'agisse de l'État, des régions, dans le cadre des CPER, ou encore de SNCF Réseau. L'entreprise s'est d'ailleurs engagée à reprendre à sa charge les investissements sur dix lignes considérées comme essentielles, lignes qui nécessitent souvent les investissements les plus importants, ce qui représente un effort très considérable de la part du gestionnaire d'infrastructures. Par ailleurs, en bonne intelligence avec les instances régionales spécialisées, une structure nationale de gouvernance va être mise en place cette année pour assurer la cohérence des volets investissements, offre de services et et innovation technique. Vous pouvez donc constater, monsieur le sénateur, que les conditions sont bien réunies pour que l'État, les régions et SNCF Réseau s'engagent sur le long terme pour la pérennité des petites lignes, à commencer par le prochain volet mobilité des CPER 2023-2027, dont l'élaboration est devant nous. La parole est

des territoires. Malheureusement, elle ne comporte pas le volet financier escompté pour les zones peu denses, pour lesquelles le versement transport reste insuffisant et devrait faire l'objet d'une péréquation nationale. Cette grave lacune a jeté la ruralité dans un dilemme cornélien : laisser la compétence aux régions et s'en remettre à leur bon vouloir, ou bien prendre une autonomie illusoire, faute de moyens,

grâce à un texte non daté, que je qualifierais d'apocryphe s'il ne figurait pas sur le site Mobilités du ministère des transports,

Confirmez-vous la validité de ce texte ministériel d'un genre nouveau, que j'ai d'ailleurs transmis à vos services ? Doit-il être colporté d'élu à élu ou allez-vous le communiquer par circulaire à tous les préfets, afin de mettre fin à cette situation d'ici au 31 mars ? Enfin, le délai ainsi obtenu sera-t-il mis à profit pour préparer le volet financier, tant attendu ?

les territoires dans la mise en oeuvre de cette loi, car ils en seront des acteurs clés. Les principaux éléments de cette note ont été rappelés le 10 février dernier par la ministre Jacqueline Gourault et par le ministre délégué Jean-Baptiste Djebbari

la note clarifie bien ce que la loi prévoit : le transfert de ces services n'est pas automatique, il est convenu entre les collectivités, uniquement sur demande de la communauté de communes. Il sera par ailleurs possible de prendre la compétence AOM sans reprendre les services régionaux internes au territoire. C'est très important. Je vous confirme donc que cette note ne déroge pas à la loi qui a été votée par

Ce projet d'aménagement du territoire vise à relier le Grand Centre et l'Auvergne au réseau européen. En attendant que ce projet se fasse, j'ai mené une enquête sur la mobilité dans un grand bassin de vie comprenant trois départements ruraux, donc peu denses : le Cher, l'Indre et l'Allier. Les premiers résultats de l'enquête ont révélé une importante attente en matière de ferroviaire, notamment dans les secteurs les plus éloignés.

Les habitants des zones rurales ne veulent pas seulement des trains, ils souhaitent qu'une articulation multimodale soit mise en oeuvre. Cela passe par une modernisation des lignes existantes, le réemploi des plus petites lignes fermées voilà quelques années et une meilleure desserte ferroviaire, à la fois d'un point de vue géographique et en termes d'horaires adaptés, ce qui n'est pas souvent le cas dans les territoires ruraux.

a enfin été entendue. Après des décennies de sous-investissement dans les lignes de desserte fine du territoire, le Gouvernement a engagé avec les régions et SNCF Réseau un plan de revitalisation comprenant plusieurs outils. D'abord, l'État, SNCF Réseau et les régions élaborent, en lien avec les contrats de plan État-région, des protocoles d'accord répartissant le financement des remises à niveau de ces lignes. Au total 7,7 milliards d'euros seront investis d'ici à 2032 pour la régénération. en réponse à une forte demande des territoires, un décret d'application de la loi LOM, publié à la fin du mois de décembre, autorise les transferts de gestion aux régions volontaires. Il leur permet d'adapter la gestion des lignes pour maintenir ou réinstaurer un service ferroviaire sur leur territoire. Par ailleurs, des études sont menées sur le développement de trains que je qualifierais de frugaux-modulables, qui permettent de réduire

Beaucoup de nos concitoyens habitant à la campagne n'ont aujourd'hui d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Leur dépendance à la voiture s'est même accrue ces dernières années avec la diminution de l'offre ferroviaire et de cars. D'autres sont contraints, faute de transport public, de renoncer à des emplois, souvent éloignés de leur domicile, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule. À cela s'ajoute une facture de carburant devenue insoutenable pour toute une partie de la France périphérique, celle qui, il y a quelques mois encore, était dans la rue en gilet jaune. Nous ne réussirons à relever le défi des mobilités en milieu rural qu'en y consacrant des moyens massifs et en en faisant une véritable priorité politique. On ne peut donc que regretter que la question de la mobilité soit traitée avec tant de légèreté dans le projet de loi Climat, ou en tout cas uniquement sous l'angle de la coercition. Promouvoir la voiture propre, c'est bien ; donner à chaque Français le même droit à la mobilité partout où il se trouve, c'est mieux ! Dès lors, comment inciter les collectivités locales à lancer des plans de mobilité ambitieux quand on sait que leurs finances sont exsangues ? Comment encourager la voiture partagée dans un contexte sanitaire qui rend les Français réticents à cette pratique ? Comment promouvoir le véhicule électrique alors qu'il reste inabordable et souvent inadapté pour beaucoup de Français vivant en zone rurale ?

La voiture individuelle est prédominante dans les territoires ruraux où, comme cela est rappelé dans le rapport, elle représentait 80 % des déplacements du quotidien en 2018. Rendre le permis de conduire plus accessible facilite l'accès à l'emploi.

Les collectivités territoriales sont le point d'ancrage du déploiement de la mobilité inclusive et solidaire dans les zones rurales. Le site internet « Tous Mobiles » a récemment été lancé avec le soutien du ministère de la transition écologique. Il propose une palette complète d'outils aux élus locaux afin de favoriser le recours au covoiturage, mais également à l'autopartage, madame la sénatrice. Je rappelle en effet que la communauté de communes de la Champagne picarde a été lauréate France Mobilités dès 2019. Son projet favorise la connaissance et l'assimilation par la population et les acteurs économiques des usages alternatifs à la voiture individuelle et des possibilités de rationaliser son utilisation à travers la promotion du télétravail, du covoiturage, de l'autostop organisé et de l'écomobilité des scolaires. Nous voulons également que les employeurs s'emparent pleinement des enjeux de mobilité. Ils y contribuent financièrement avec le versement mobilité pour les services réguliers et peuvent désormais contribuer aux déplacements à vélo ou en covoiturage de leurs salariés. Si le Gouvernement est aussi proactif et favorise l'émergence de solutions de mobilité partout et pour tous, c'est justement parce qu'il est insupportable, vous avez raison, qu'un Français sur quatre soit obligé de refuser un emploi, faute d'accès à une offre de mobilité adaptée. Pour finir, je vous indique que le projet de loi Climat et résilience, dont l'Assemblée nationale est saisie, comprend un titre III intitulé : « Se déplacer ». Il vise justement à promouvoir les mobilités alternatives à la voiture individuelle.

Le sujet des mobilités est en effet majeur pour nos territoires, où se déplacer est parfois compliqué, souvent coûteux, de le dire Pascale Gruny à l'instant, mais toujours nécessaire. Nous le savons, les mobilités sont en pleine évolution, mais le constat est là : c'est dans les grandes agglomérations que les transformations ont lieu. Les espaces ruraux restent, pour l'essentiel, à l'écart de ce mouvement. C'est bien cela qui nous inquiète. Plus les évolutions seront rapides, plus l'écart se creusera entre, d'un côté, les territoires où se déploieront une palette d'offres intéressantes et les innovations technologiques les plus abouties et, de l'autre, des territoires moins peuplés, au relief plus compliqué- c'est un élément important -, qui se sentiront de plus en plus éloignés du progrès et délaissés par ceux qui mettront en place les nouveaux services. Devoir continuer à dépendre uniquement de sa voiture individuelle pendant que toutes sortes de modes de transports alternatifs et socialisés se mettent en place dans les villes contribuera malheureusement à accroître le sentiment de relégation que connaissent un certain nombre de nos concitoyens dans les territoires ruraux. C'est pourquoi une attention particulière doit leur être portée. Je retiens de ce débat que, pour préparer l'avenir, nous devrons prendre en compte trois contraintes. La première est bien sûr la contrainte écologique.

innovations dans le domaine des mobilités reposent sur le numérique, nous l'avons mesuré ce soir. Il est donc impératif que la couverture numérique de notre territoire soit complète. Soyez assurés que l'Ardéchois qui vous parle mesure jour après jour le chemin qu'il reste à parcourir. La troisième est la contrainte organisationnelle. La LOM prévoit que tout le territoire sera couvert par une autorité organisatrice de la mobilité à compter du 1 juillet prochain. C'est une chance pour permettre la conception de services adaptés aux spécificités des territoires- de tous les territoires. Encore faut-il que les acteurs locaux s'en saisissent pleinement et soient accompagnés. Des moyens humains, financiers, d'ingénierie territoriale

dans les espaces peu denses. Pour ma part, j'en tire trois conclusions. La première est que le n'est pas possible. Il ferait même peser un risque certain sur l'attractivité des territoires concernés. La deuxième est est qu'offrir une palette de solutions variées et adaptées doit être l'ambition des acteurs territoriaux de la mobilité. L'avenir reposera assurément, de plus en plus, sur des offres multiples, conçues au plus près

Que ce soit dans un cadre professionnel ou associatif, organisé ou spontané, expérimental ou en voie de régulation, l'appropriation des outils des mobilités partagées est une réalité sur laquelle nous pourrons miser. Comme le disait Pierre Massé, grand commissaire au Plan, « Le regard sur l'avenir est le premier temps de l'action ». C'est pourquoi la délégation à la prospective a voulu que ce débat ait lieu ce soir. Nous sommes convaincus, que c'est bien dès aujourd'hui que l'on doit commencer à préparer l'avenir des mobilités dans nos campagnes. Nous espérons que vous aurez entendu ce message, monsieur le secrétaire d'État. La délégation La délégation à la prospective continuera de porter son regard sur l'avenir, de réfléchir aux transformations de la société et de l'économie, pour, conformément à sa mission, en informer le Sénat. Mes chers

La séance est levée.